citoyen et écologiste. Madame la ministre, après deux semaines de grèves et de manifestations, notamment celle d'hier, à l'appel de toutes les organisations syndicales, après les scandales qui ont éclaboussé votre ancien et éphémère secrétaire d'État, vous continuez à défendre l'indéfendable, en répétant que tout le monde sera gagnant avec votre projet de réforme des retraites. dans tous les pays où le système de retraite par points a été mis en oeuvre, l'ensemble du monde du travail a dû travailler plus longtemps pour gagner moins. Vous essayez de monter les Françaises et les Français les uns contre les autres- régimes spéciaux contre régime général, jeunes contre vieux -, mais tout le monde a bien compris que votre pseudo-régime universel était une machine à fabriquer précarité et misère sociale. Les manifestantes et manifestants d'hier sont autant de porte-voix pour démonter votre entreprise d'intox et d'enfumage, comme les associations féministes et les syndicalistes réunis lundi soir à la Maison des métallos pour s'élever contre votre argumentaire, selon lequel les femmes seront les grandes gagnantes, quand elles sont les premières perdantes. Madame la ministre, la France est dans la rue, personne ne veut de votre néfaste projet, à part vos amis du Medef et de la haute finance. Ma question est simple : quand allez-vous retirer votre réforme ?

de solidarité intergénérationnelle. Le système n'est plus adapté aux changements de métier. Il pénalise les personnes qui passent d'un statut à un autre. C'est un système fondé sur les statuts, et non sur les trajectoires individuelles de chacun de nos compatriotes. Il ne

la nomination du nouveau « M. Retraites », qui a à son actif le licenciement d'une caissière d'Auchan pour quelques centimes d'euros, est loin d'apaiser l'inquiétude et la colère dans le pays. Contrairement à ce que vous dites, les mobilisations sont largement soutenues par les Françaises et les Français, qui ne veulent sacrifier ni leurs vieux jours ni ceux de leurs enfants. Quant à vos arguments comptables, ils sont nuls et non avenus. Le « pognon de dingue » existe : c'est l'explosion des revenus du capital, qui ne participe pas au financement des retraites.

SMIC. Nous avons un point d'accord : nous avons le meilleur système de retraites du monde. Il est encore perfectible, mais son financement serait assuré sur le long terme si vous cessiez d'y puiser. Vous avez résolu de casser le système plutôt que de l'améliorer, avec pour conséquences inquiétudes, injustices et pauvreté, sans garantie réelle sur la valeur du point, sans précisions sur les 12 milliards d'euros pour les enseignants, sans correctifs pour les carrières erratiques des jeunes, les 900 000 chômeurs que vous allez fabriquer ou encore les carrières interrompues et des pensions de réversion à 62 ans au lieu de 55- j'en oublie ... L'âge pivot, lui,

Vous exhortez à une trêve sans la souhaiter vraiment. En effet, quel geste faites-vous ? Il suffirait d'abandonner dès aujourd'hui la référence inopportune et punitive à l'âge pivot, de remettre sur le métier votre ouvrage, de le reprendre totalement, sans dogme sur le système, de parler vrai, d'associer les corps intermédiaires, d'écouter la population pour présenter un projet de justice et d'avenir, un projet digne de confiance- confiance que vous avez érodée et que bien peu vous accordent encore. Y êtes-vous prêts ?

d'urgence se déclenche dans nos rues ? En 2013, cette question a été posée aux Français : 78 % d'entre eux ne le savaient pas.

sur un périmètre prédéfini, en les alertant individuellement, non seulement sur le phénomène qui vient de se produire et dont elles doivent se préserver, mais également sur les mesures à prendre.

par message électronique. Les pouvoirs publics pourront s'adresser aux opérateurs de téléphonie mobile pour diffuser ces messages. Mais le plus important, comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur,

qui allaient conduire à une grave crise du logement et du bâtiment en 2021. Je ne m'étais pas trompé, monsieur le ministre : en cette fin d'année, le marché du logement neuf est durablement affecté. Le nombre de logements offerts à la vente baisse de 14 %. Le stock est inférieur à neuf mois. La délivrance des permis de construire dans le logement collectif chute de 25 %. En conséquence, les prix augmentent de 4,7 %. La Fédération des promoteurs immobiliers parle d'un immense gâchis.

Pour ce qui concerne l'accession à la propriété, la fin programmée du prêt à taux zéro (PTZ) sous sa forme actuelle, provisoirement sauvé par la majorité sénatoriale, entraînera une nouvelle baisse de la construction. Si vous ne changez rien, nous aurons mécaniquement perdu 50 000 constructions en trois ans.

un décrochage de la construction. On n'attend pas plus de 385 000 mises en chantier en 2021. Du temps du plan Borloo, que j'ai eu l'honneur de mettre en oeuvre, il y en avait 490 000 ! Or 100 000 constructions de moins, c'est 250 000 emplois de moins dans le bâtiment. Monsieur le envisagez-vous un plan de relance pour faire face à ce problème, comme nous l'avons fait avec succès en 2008 les chiffres que vous venez d'évoquer ne sont évidemment pas satisfaisants. Aujourd'hui, il faut accroître les efforts pour relancer la construction. En 2018, on dénombrait environ 420 000

et a menacé de récidiver durant les fêtes. Une telle attitude est inacceptable et nous la condamnons vivement. Près de 170 000 foyers, des quartiers entiers, ont été impactés dans toute la France : 40 000 à Lyon, 40 000 à Orléans et à Nantes et près de 50 000 dans mon département de la Gironde. Au-delà des particuliers, ce sont aussi des services publics indispensables qui ont parfois été bloqués, comme des crèches, des hôpitaux ou des services administratifs. Je pense aussi aux commerçants, qui subissent une double peine, après les manifestations des « gilets jaunes outre la gêne qu'elles occasionnent, ces coupures sont manifestement illégales. La direction de RTE a annoncé que des plaintes avaient été déposées et que des sanctions disciplinaires seraient mises en oeuvre. Pour autant, le syndicat semble indiquer qu'il n'hésiterait pas à reconduire des actions du même type, en agitant la menace de coupures plus importantes. Madame la ministre, mes questions sont très simples : quelles actions le Gouvernement compte-t-il entreprendre afin que ces actes soient non seulement condamnés, mais également empêchés ?

Les conséquences de ces actes pourraient être dramatiques. Ce n'est pas admissible. Je condamne donc avec la plus grande fermeté les coupures d'électricité volontaires survenues ces dernières heures sur le réseau électrique.

grévistes, qui ne sont pas toujours salariés des opérateurs eux-mêmes et que je ne confonds pas avec l'immense majorité des agents du service public, qui sont attachés à leur mission.

définie comme le fait de consacrer plus de 8 % de ses revenus pour régler la facture énergétique de son logement, touche en moyenne près d'un Français sur huit. À l'échelle francilienne, les chiffres sont encore plus dramatiques : selon le baromètre Qualitel, près de 60 % des Parisiens déclarent avoir « souvent » ou « parfois » froid dans leur logement, soit 12 points de plus que la moyenne nationale. Il s'agit là d'un enjeu prioritaire, auquel le Gouvernement ne peut et ne doit pas rester sourd, car il frappe tout particulièrement les foyers les plus modestes. Lorsqu'ils cherchent à améliorer le confort thermique de leur logement, en engageant, par exemple, des travaux d'isolation ou de changement de chaudière, les ménages souffrent notamment d'un manque inquiétant d'information et de lisibilité sur les dispositifs d'aide existants.

Mes questions sont les suivantes : où en est-on, madame la secrétaire d'État, du déploiement de ce programme ? Quelles sont les régions qui sont dès à présent prêtes à contractualiser avec l'État dans ce domaine ? Enfin, quels sont les autres moyens déployés par le Gouvernement pour répondre à ce fléau qu'est la précarité énergétique ? La parole

les certificats d'économies d'énergie, pour contractualiser sur trois ans afin d'assurer un service neutre et gratuit à la totalité de nos concitoyens.

Monsieur le secrétaire d'État, ce lundi 16 décembre, votre ministère a annoncé que le vaccin contre le papillomavirus (HPV) sera désormais recommandé pour les garçons de 11 ans à 14 ans, au même titre que pour les jeunes filles. C'est pour nous une excellente nouvelle. Les bénéfices de la vaccination généralisée des adolescents sur la réduction du nombre des cancers génitaux et oraux déclarés à l'âge adulte ne sont plus à démontrer. Plus de 6 000 nouveaux cas de cancers liés aux infections par le papillomavirus sont détectés chaque année en France, dont un quart chez les hommes. Oui, les hommes sont aussi concernés : ils peuvent être porteurs du virus et le transmettre et sont aussi susceptibles de déclarer un cancer de l'appareil génital ou de la sphère ORL.

efficace existe. Or notre couverture vaccinale est l'une des plus faibles d'Europe et peine à dépasser 20 %. Dans d'autres pays, le virus est sur le point d'être éradiqué. En Australie, par exemple, la campagne de vaccination gratuite des adolescents a produit des résultats spectaculaires la proportion des jeunes femmes porteuses a chuté de 23 % à 1 % en à peine dix ans. Monsieur le secrétaire d'État, il faut à tout prix casser la chaîne de cette contamination. Une première étape a été franchie avec l'expérimentation, en Guyane et en Grand Est, de la vaccination des jeunes filles en milieu scolaire. Je salue cette initiative. voilà peu de temps, une fédération de parents d'élèves a fait circuler dans ma région une lettre dénonçant « une décision politique autoritaire d'une extrême gravité » et a introduit ainsi le doute, et encore le doute. Monsieur le secrétaire d'État, comment allez-vous répondre aux inquiétudes de certains parents et faire face aux désinformations mortifères de certains groupuscules ? Pouvez-vous nous préciser si le vaccin contre le HPV sera remboursé pour les garçons ? Ne pensez-vous pas que son ajout à la liste des onze vaccins obligatoires est enfin nécessaire ?

et de la santé, que cette recommandation soit intégrée dans le calendrier des vaccinations de 2020, pour une mise en oeuvre d'ici à l'été prochain. La vaccination étendue à tous les jeunes garçons est une décision à la fois scientifique et éthique qui leur permettra, quelle que soit leur orientation sexuelle, de bénéficier d'une protection individuelle, mais aussi, comme pour la vaccination des jeunes filles, d'améliorer la protection de leur partenaire. Cette vaccination, associée au dépistage du cancer du col de l'utérus, constitue la meilleure stratégie de lutte contre ce cancer qui provoque en France, vous l'avez rappelé, madame la sénatrice, près de 1 000 décès par an chez les femmes. Soyez convaincue, et la démonstration n'est plus à faire, de l'engagement de la ministre des solidarités et de la santé en faveur de la politique vaccinale et de la couverture vaccinale dans notre pays. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, quelle déception ! Quatre ans après l'accord historique de Paris qui avait suscité tant d'espoir et d'enthousiasme, la COP25 s'achève sur des décisions insignifiantes. Échec à relever l'ambition et à réglementer les marchés du carbone, fiasco annoncé du mécanisme des pertes et préjudices envers les pays en voie de développement ... Aujourd'hui, l'inaction des États est pointée du doigt et creuse le fossé démocratique entre les dirigeants et les aspirations citoyennes. Où se situe notre crédibilité quand notre président, pourtant sacré champion du monde, est aux abonnés absents ? C'est un lourd manquement politique à la cause climatique. Quelle ironie, d'ailleurs, quand le stand de la France à Madrid affichait sur un écran lumineux, de manière décalée, quasi surréaliste : « Mobilisation générale », comme une radicalité désincarnée de dernière chance. Les générations futures sont dans la rue et nous interpellent face à une promesse d'avenir qui s'efface fonte du pergélisol, progression des déserts, canicules à répétition, baisse drastique de la biodiversité ... Les objectifs dérapent sur l'impossibilité d'intégrer dans notre société la réalité du changement climatique.

qu'en 2040 à nouveau ... Le mot urgence a-t-il pour vous un sens ? Notre modèle de consommation est dépassé, nous l'avons épuisé. Nous allons de reculade en reculade et le temps des grands-messes inopérantes devrait être derrière nous. Quand assumerez-vous votre rôle ? La parole est à

oui, alors que l'urgence climatique est là, alors que les citoyens se mobilisent partout dans le monde, l'ambition a manqué à cette COP25 et la France le regrette vivement. Je voudrais remercier la présidence chilienne de cette COP et l'Espagne, pays d'accueil, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que cette rencontre internationale sur le climat puisse produire des effets. Durant deux semaines, la France s'est mobilisée comme peu de pays l'ont fait, avec l'Union européenne, avec nos partenaires, pour ne pas accepter le recul des engagements des accords de Paris et pour appeler à l'action en vue de la COP26, à Glasgow. Le Premier ministre s'est rendu avec Brune Poirson à l'ouverture de cette COP et Élisabeth Borne y était également, dans dans le segment ministériel, pour les négociations sur l'accord de clôture. Le résultat est certes décevant, j'en conviens. Cette COP a néanmoins permis d'acter certaines avancées utiles à la mise en oeuvre des accords de Paris. Je pense, par exemple, à la création d'un groupe de travail sur l'accompagnement des pays vulnérables dès 2020, à la mobilisation du réseau de Santiago pour faciliter les collaborations face aux risques naturels ou à la création d'un nouveau fonds fiduciaire consacré à la biodiversité. Nous devons continuer de travailler, notamment avec nos partenaires de l'Union européenne, pour adopter le plus rapidement possible un objectif rehaussé de réduction de nos émissions d'ici à 2030. C'est l'un des enjeux de la prochaine COP.

Le monde craque sur l'inefficacité des politiques. Il est grand temps de considérer la nature comme un capital gratuit, mais sans garantie. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, en ce quatorzième jour de grève contre la réforme des retraites, les chambres de commerce et d'industrie (CCI) commencent à publier leurs premières statistiques mesurant l'impact économique de ce mouvement social sur les commerces et les entreprises. Comme nous pouvions l'anticiper, c'est en région parisienne, là où la grève dans les transports pose le plus de problèmes et concerne le plus grand nombre de nos compatriotes, que les conséquences économiques sont les plus lourdes. Les pertes d'activité déclarées par les professionnels sont importantes. Elles auront, dans les semaines et les mois à venir, des conséquences sociales avec leur inévitable lot de cessations d'activité et de placements en chômage partiel, voire définitif. Alors que le mois de décembre et la fin d'année représentent souvent une part importante du volume d'affaires de beaucoup de commerces parisiens, les chiffres de cette première moitié du mois sont inquiétants : baisse de 80 % pour les commerces situés dans les gares ou à proximité,

En moyenne, près des deux tiers des artisans ou commerçants franciliens se déclarent impactés ! Madame la secrétaire d'État, que prévoyez-vous pour aider les entreprises qui vont se retrouver en difficulté, au-delà du désormais traditionnel étalement des impôts et cotisations sociales ?

comme vous le savez, depuis le 5 décembre dernier, le ministre de l'économie et des finances et moi-même faisons le point tous les deux jours avec les fédérations et les chambres consulaires pour prendre la mesure de l'impact des blocages que nous subissons en ce moment, essentiellement en Île-de-France, comme vous l'avez souligné, sur le commerce et l'artisanat.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le feuilleton de la consigne n'en finira donc jamais. Alors que le Sénat avait clarifié le dispositif flou de la consigne en le recentrant sur le réemploi, alors que le Gouvernement s'est engagé à une concertation étroite avec les élus locaux et que le président de la République a affirmé que rien ne se ferait sans l'accord des maires, alors que votre gouvernement défend, d'une part, la protection de l'environnement et, d'autre part, la capacité de différenciation des collectivités territoriales,

Cet accord aurait permis d'expérimenter des dispositifs de consigne territoriale dès 2020, de faire un point d'étape en 2025 sur les capacités de récupération des bouteilles en plastique au regard de nos engagements européens et d'envisager un dispositif de consigne si la trajectoire des 90 % de collecte en 2029 ne semblait pas respectée. Madame la secrétaire d'État, le geste de tri est ancré dans le comportement de nos concitoyens.

de la transition écologique et solidaire. Monsieur le sénateur Longeot, une concertation a lieu depuis plusieurs mois sur la question de la mise en oeuvre de la consigne. Comme le Président de la République et le Premier ministre l'ont rappelé à l'occasion du congrès des maires, rien ne pourra être fait sans les associations de collectivités territoriales qui sont chargées du service public de gestion des déchets et de la propreté. C'est dans cet esprit qu'Élisabeth Borne et Brune Poirson ont trouvé un accord avec les associations de collectivités, le 25 novembre dernier

L'amendement du Gouvernement sur la consigne reprend point par point l'accord trouvé entre Élisabeth Borne, Brune Poirson et les associations d'élus. Cet accord est respectueux des objectifs écologiques voulus par le Gouvernement et la majorité et des intérêts des collectivités locales. Nous souhaitons avancer avec l'ensemble des acteurs locaux, raison pour laquelle cet amendement vise à lancer des expérimentations de consignes mixtes pour recyclage et pour réemploi sur les territoires volontaires, par exemple en outre-mer, et à généraliser, au terme d'un bilan d'étape en 2023, notamment sur l'atteinte des objectifs de collecte des plastiques par les collectivités, après concertation après concertation avec les collectivités, des systèmes de consignes mixtes pour recyclage du plastique et pour réemploi du verre sur tout le territoire. Les collectivités ont dénoncé hier l'accord qu'elles avaient validé et souhaitent ajouter de nouvelles conditions qui conduiraient, si elles étaient votées, à ce que la consigne ne puisse jamais voir le jour en France. L'amendement actuellement défendu à l'Assemblée nationale est le fruit d'un compromis. Nous espérons vivement que chacun aura à coeur d'être responsable pour avancer ensemble sur ce sujet.

Défendre, aider le patrimoine en France est devenu une urgence. Le patrimoine touche à ce que nous sommes. Comme M. Riester l'a justement dit, « ce n'est pas seulement ce que nous recevons ; c'est aussi ce que nous transmettons Le loto du patrimoine est un succès populaire. Preuve, s'il en était besoin, que les Français sont attachés à leur patrimoine. Et lorsqu'ils jouent au loto, c'est avec la conviction profonde que les sommes qu'ils dépensent vont au patrimoine et ne remplissent pas le puits sans fond de Bercy. Afin de ne pas tricher avec les Français, le Sénat a adopté, le mois dernier, une disposition de bon sens visant à affecter la totalité des sommes prélevées à la sauvegarde de notre patrimoine.

C'est méconnaître l'importance du patrimoine, facteur d'attractivité des territoires, de développement local et de cohésion sociale qui attire, je vous le rappelle, 90 millions de visiteurs chaque année et impacte la vie de 500 000 salariés. Comprenez-vous, madame la secrétaire d'État, la colère de Stéphane Bern ? Êtes-vous favorable au retour de la taxe défendue par le tout-puissant, je dirais même le trop puissant, ministère des finances ?

Comme vous l'avez rappelé, le loto du patrimoine est un grand succès populaire qui a permis de mobiliser les Français autour de notre patrimoine, en particulier autour de notre petit patrimoine. Il a dégagé plus de 22 millions d'euros de recettes en 2018

de taxes ! Répondez ! De surcroît, en 2018, l'État a accompagné pleinement cette mobilisation populaire à travers un dégel de la réserve du programme « Patrimoine » ... Je trouve assez cocasse que ce soit sur les travées de la droite qu'on nous reproche d'être soucieux des deniers publics en utilisant l'arme du gel Cet engagement du Gouvernement a été maintenu pour la seconde édition et nous nous en félicitons. Comme en 2019, ces moyens supplémentaires seront intégralement consacrés, en 2020, à abonder, via les directions régionales des affaires en péril à hauteur des taxes du loto. Ce financement permet ainsi à l'État de compléter les moyens déjà consacrés aux travaux des monuments en péril au taux maximum possible. Cet effort budgétaire significatif exceptionnel permet ainsi de mobiliser véritablement des fonds supplémentaires en faveur de la restauration du patrimoine. Je veux également rappeler l'effort du ministère de la culture en matière de monuments historiques qui s'élèvera, l'an prochain,

Il s'appelait Jess, il avait 17 ans. Il était sous la protection de l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Hauts-de-Seine. Mercredi dernier, nous avons appris avec tristesse et colère la mort de ce jeune, poignardé par un autre jeune de 15 ans, lui aussi placé. Ce drame s'est déroulé dans un hôtel de Suresnes qui accueille des populations fragiles, souvent placées par le 115. Un hôtel, monsieur le secrétaire d'État, où étaient hébergés trente enfants, « faute de mieux

Les travailleurs sociaux, les personnels de l'ASE, sont souvent le seul lien qui reste pour ces jeunes. Dès lors, comment accepter qu'ils aient sous leur responsabilité entre soixante Désespérés, ils nous avaient alertés : « Si cette inaction perdure, un drame va se produire. » Ce drame est arrivé. Nous le savons, monsieur le secrétaire d'État, la plupart des départements mènent une politique volontariste, malgré des contraintes économiques importantes, et nous devons les accompagner davantage. Mais, dans le même temps, d'autres départements enregistrent des excédents budgétaires faramineux et continuent de fermer des structures, de supprimer des postes et abandonnent les enfants sous leur protection, relégués à n'être que de simples variables d'ajustement budgétaire. des affaires sociales (IGAS) de mener une mission de contrôle de l'aide sociale à l'enfance dans les Hauts-de-Seine et de dresser un état des lieux complet au niveau national sur la question de l'hébergement. Je tiens à saluer cette initiative. Monsieur le secrétaire d'État, le plan que vous avez présenté le 14 octobre dernier permettra- je le souhaite -d'améliorer la prise en charge des enfants placés. Mais nous ne pouvons plus accepter l'inaction de certains, qui, par choix politique, refusent délibérément de prendre leurs responsabilités.

le Gouvernement s'est engagé, comme nous tous ici, à améliorer les conditions d'accueil et d'accompagnement des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. C'est la raison pour laquelle, avec Agnès Buzyn, nous avons saisi l'IGAS pour qu'elle mène une mission de contrôle sur l'aide sociale à l'enfance dans les Hauts-de-Seine, afin d'améliorer la prise en charge de ces enfants, et qu'elle réalise un audit complet, sans fard, sur les conditions de prise en charge des enfants dans des lieux non autorisés sur l'ensemble du territoire national. Les recommandations de l'inspection générale des affaires sociales viendront utilement alimenter les travaux que nous avons déjà menés dans le cadre de la stratégie que j'ai présentée le 14 octobre dernier et qui vise à améliorer, à mieux encadrer, à mieux normer les conditions d'accueil et d'hébergement des enfants dans notre pays au sein de structures autorisées. Plus largement, vous pouvez compter sur le Gouvernement, et je sais pouvoir compter sur vous, pour aller dans ce sens. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Ma question s'adresse à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire. Les études scientifiques sur la fonte des glaciers et la disparition des espèces ne se comptent plus tant elles sont nombreuses. Les préoccupations des Français, notamment des plus jeunes, concernant l'état de notre environnement et l'urgence climatique sont de plus en plus importantes. Les citoyens attendent une forte mobilisation des politiques pour nous adapter au changement climatique et préserver notre biodiversité. Sur le terrain, les collectivités locales en ont pris conscience et sont de plus en plus engagées. Les grandes conférences internationales que sont les COP sont certainement nécessaires pour impulser une mobilisation mondiale et sensibiliser les États. Encore faut-il qu'elles soient réellement utiles et aboutissent à du concret. La COP25 de Madrid, la COP la plus longue de l'histoire, est apparue comme déconnectée par rapport aux demandes d'action exprimées. Les résultats sont consternants tant ils sont faibles. Les négociateurs n'ont pas pu s'entendre sur les règles d'application de l'accord de Paris concernant la question clé du marché carbone. Aucun État ne s'est engagé pour participer au fonds vert. La question des « pertes et préjudices », à savoir les destructions déjà irréversibles liées au réchauffement, notamment en Afrique, avec la création d'un fonds, un échec. Ce n'est pas possible ! On risque de décrédibiliser définitivement les sommets internationaux. Cette COP avait besoin d'un leadership politique. Où est passé le leadership français,

face à la transition écologique qui est devant nous, que ce soit en termes de lutte contre le réchauffement climatique ou de lutte contre la perte de biodiversité. Pourtant, la France a été l'un des États qui s'est le plus mobilisé dans cette COP, avec la visite du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, et de Brune Poirson, secrétaire d'État chargée du dossier, pour participer aux négociations. Nous avons oeuvré pour obtenir des avancées. Je pense, par exemple, à la reconnaissance de la science et des rapports du GIEC par cette COP, reconnaissance qui était loin d'être acquise si l'on considère le scepticisme de certains États. Surtout, cette COP a été l'occasion d'avancer au niveau européen. Le Conseil européen qui s'est tenu à la même période a validé l'objectif de la neutralité carbone à l'échelle de l'Union européenne en 2050, avec un accord de tous les États membres, sauf de la Pologne- elle continue à y travailler -, ce qui nous permettra de transposer cette volonté, déjà à l'adoption de la loi Énergie-climat, à l'échelle européenne. Nous travaillons également sur le rehaussement des objectifs à l'horizon de 2030 et sur le mécanisme de compensation, souhaité depuis longtemps

dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'action doit être internationale, nationale et locale. C'est la raison pour laquelle je porte, pour ma part, 80 contrats de transition écologique locaux, auxquels nous travaillons avec toutes les collectivités locales, pour que l'écologie s'inscrive, concrètement, dans le quotidien des Français. La parole est pour la réplique. Madame la secrétaire d'État, j'entends votre réponse. Toutefois, on ne peut que s'étonner de l'absence du Président de la République à la COP, alors même qu'il se targue de mettre l'environnement au coeur de l'acte II du quinquennat. Quelle est l'authenticité de l'engagement de l'exécutif ?

Nous sommes au bord du drame. L'hôpital public se meurt ». C'est ainsi que débute la tribune publiée il y a quelques jours par 660 médecins hospitaliers, lesquels, s'adressant au Gouvernement, affirment envisager de démissionner s'ils ne sont pas écoutés. À Marseille, le service de réanimation pédiatrique fait face à une épidémie, avec 20 % de ses lits fermés et 12 infirmières manquantes. Des assignations sont adressées aux internes pour tenter de maintenir tant bien que mal la permanence des soins. Au CHU de Toulouse, 243 signalements révélant de graves dysfonctionnements ont été recensés en une année. L'établissement est au bord de l'implosion. À l'AP-HP, il y avait 400 postes d'infirmières vacants en septembre. Il y en a 692 cette semaine. Dans de nombreux territoires, de telles situations se répètent ; elles inquiètent nos concitoyens et nous tous, ici, sur ces travées. Madame la ministre, la situation continue de s'aggraver malgré vos annonces successives. Quand comptez-vous apporter des réponses à la hauteur de la crise, celle d'un affaissement, que vit l'hôpital public dans nos territoires ?

Malheureusement, quand le chef de l'État a lancé le grand débat national, il a oublié la santé. Les Français lui ont répondu en la mettant au premier rang de leurs préoccupations. Il faut enfin débattre ensemble de la place de l'hôpital public et des moyens qu'on lui consacre.

après Julien Denormandie pour l'habitat, Jean-Michel Blanquer pour les écoles, c'est accompagné de Mme Belloubet et de M. Darmanin que vous êtes venu, monsieur le ministre, au mois de septembre. Il ne manquait plus à cette caravane humanitaire que Bernard Kouchner avec son sac de riz sur le dos Votre venue dans notre belle cité phocéenne était motivée par la présentation en grande pompe de votre plan antidrogue. Les caméras éteintes, vous êtes rentré à Paris, et la vie, ou plutôt la mort, a repris ses droits, avec deux nouvelles victimes à l'occasion de règlements de compte.

ou même La Poste, les télécoms ou EDF, voire d'interroger le boulanger du coin- s'il n'a pas fui -, pour constater que tout le monde connaît les points de deals et même le nom des trafiquants. Marseille est gangrénée par les mafias. Elles ont contaminé des pans entiers de l'économie légale. L'argent abondant et facile aveugle des gamins, dont beaucoup trop de mères finissent par verser des larmes de sang. Des cités entières sont sous la coupe de crapules, et ce sont les honnêtes gens, prisonniers des trafics, qui se retrouvent cloîtrés, barricadés, incarcérés chez eux ! Pour s'attaquer au deal, il faut s'attaquer à l'argent qu'il génère. Il faut mettre les trafiquants sur la paille, en les empêchant de bénéficier du fruit pourri de leur business. Combien d'entre eux sont propriétaires de restaurants toujours vides, d'épiceries de nuit toujours désertes, de kebabs ou de boutiques de téléphonie mobile, alors qu'ils ne déclarent aucun revenu ? Il est là le point sur lequel vous devez porter le fer. Monsieur le ministre, la guerre contre la drogue doit être totale. Pour la mener, les États-Unis ont mis 16 milliards de dollars sur la table en 1998, soit pas moins de 60 dollars par habitant. Votre question ! Ma question est la suivante : allez-vous enfin accorder 60 euros par Marseillais

La séance est reprise. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- vingt voix pour, sept voix contre -à la nomination de M. Pierre Dubreuil aux fonctions de directeur général de l'Office français de la biodiversité. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet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 L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l'adoption de ce texte. Je mets aux voix le texte à l'adoption de ce texte. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres,

l'examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances (PLF) constitue toujours un exercice particulier. Cette année ne fait pas exception à la règle, puisque la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à un accord sur l'ensemble des dispositions du PLF pour 2020. Je veux tout d'abord saluer l'implication de tous les sénateurs, ces dernières semaines, sur ce texte, pendant de nombreuses heures de débat. Sur les 393 articles figurant dans le texte adopté par le Sénat, 111 ont tout de même été votés conformes, soit un peu moins d'un quart. Le texte qui vous est soumis aujourd'hui a été modifié par l'Assemblée nationale. Sans surprise, le Gouvernement a d'abord souhaité rétablir les crédits des cinq missions que vous aviez rejetées : « Sécurités », « Écologie, développement et mobilité durables », « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Justice » et « Immigration, asile et intégration ». Ces annulations conduisaient à une réduction, évidemment artificielle, des dépenses de 52,7 milliards d'euros, ce qui n'est, compte tenu de l'importance de chacune de ces missions, ni souhaitable ni crédible. Le Gouvernement s'est aussi opposé à toutes les mesures qui visaient à remettre en cause les réformes que nous conduisons depuis plus de deux ans et demi. Vous le savez, nous avons un objectif de redressement de nos comptes publics.

Aussi le Gouvernement propose-t-il dans ce projet de loi de finances de poursuivre la démarche initiée l'année dernière pour réduire le nombre de dépenses fiscales inefficientes. Nous avons ainsi renouvelé notre opposition aux dispositions que vous avez adoptées et qui visaient au contraire à renforcer certaines dépenses fiscales.

bonne chose. Cela aurait réduit la lisibilité pour les contribuables et les élus des modalités de la suppression et de la compensation de la taxe d'habitation. Néanmoins, le Gouvernement s'est engagé à établir des simulations extrêmement précises, afin de s'assurer que la réforme de la fiscalité ne désorganise pas la répartition des dotations versées par l'État aux collectivités à partir de 2022, notamment au regard des potentiels fiscal et financier.

finances locales) est d'ores et déjà prévu dès la mi-janvier, pour aborder les conséquences de la réforme fiscale sur les indicateurs de ressources utilisés pour le calcul des dotations et des fonds de péréquation. Celle nouvelle lecture a été l'occasion pour le Gouvernement de tirer les conséquences de certaines annonces intervenues depuis la première lecture, notamment s'agissant du déplafonnement du malus automobile et du plan de soutien à la filière automobile. automobile. Le dispositif d'accompagnement financier des régions dans le cadre de la réforme de l'apprentissage a été également ajusté et renforcé, en rehaussant le niveau des ressources qui leur sont affectées à l'article 24. Ce point avait été soulevé par M. Bruno Retailleau. Nous avons trouvé une solution, grâce à un soutien supplémentaire à l'apprentissage à hauteur de 50 millions d'euros, en sus des 228 millions d'euros déjà prévus dans le projet de loi de finances, comme le Gouvernement s'y était engagé ici même. même. L'État et France compétences verseront donc environ 600 millions d'euros aux régions, tout en reprenant les charges induites. Les 50 millions d'euros supplémentaires ont été répartis au prorata des primes d'apprentissage en 2020 et 2021,

non routier), deux amendements du Gouvernement ont été adoptés par l'Assemblée nationale, afin d'accompagner les artisans des travaux publics dans le cadre de la suppression du tarif réduit du GNR. La première mesure met en oeuvre un suramortissement pour le renouvellement des engins de plus de cinq ans, afin de renouveler le parc avec des engins moins polluants. La seconde instaure un renforcement des contrôles sur le terrain, impliquant notamment une coloration spécifique de carburant pour les travaux publics et l'établissement d'une liste d'engins de chantier réputés non éligibles au tarif agricole, définie par arrêté et qui fera l'objet d'une concertation. Un renforcement des responsabilités des donneurs d'ordre est également prévu avec la création d'un registre des travaux relevant du secteur des travaux publics réalisés par les entreprises agricoles, assortie de sanctions douanières en cas de non-tenue du registre ou d'absence de mise à jour. le souligne, mesdames, messieurs les sénateurs, la sincérité de notre budget est une priorité. Cette nouvelle lecture est l'occasion d'actualiser nos prévisions de recettes et de dépenses, en cohérence avec les dernières informations qui vous ont été présentées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2019. 2019. La reprise des plus-values fiscales de l'année 2019, notamment sur les droits de mutation, nous conduit à rehausser la prévision de recettes de 1,4 milliard d'euros en 2020. Pour ce qui concerne les dépenses, au vu du dynamisme des prestations sociales observé en 2019, nous proposons d'augmenter significativement, à hauteur de 750 millions d'euros, les crédits consacrés à la prime d'activité et à l'allocation aux adultes handicapés. En tenant compte des prévisions de fin d'année dès la loi de finances initiale, dans l'objectif d'une budgétisation au plus juste des dépenses obligatoires, nous préparons une gestion plus soutenable et plus sereine. Je le répète, nous ne souhaitons pas nous trouver contraints de prendre des décrets d'avance. Ces ajustements nous conduisent à revoir très légèrement à la hausse le déficit de l'État, d'environ 93 millions d'euros. Il s'établira ainsi à un peu plus de 93 milliards d'euros, qui n'entraîne pas de modification de notre prévision du déficit public en 2022, que nous maintenons à 2,2 %. Dans la continuité de notre action depuis deux ans, nous maintenons notre exigence de discipline budgétaire. Les amendements relatifs aux crédits que nous vous soumettrons participeront ainsi de notre démarche de sincérisation des comptes.

Elle a maintenu l'exclusion du président du conseil de surveillance et du président du conseil d'administration lorsque ce dernier n'assume pas la fonction de président-directeur général. Confirmant le vote du Sénat, l'Assemblée nationale est revenue

en conservant le renforcement des clauses anti-abus adopté par le Sénat. Parmi les principaux apports, on peut également citer les modifications substantielles introduites à l'article 58 relatif à la création d'une réduction d'impôt sein des foncières solidaires, y compris son extension aux foncières solidaires à vocation agricole. L'Assemblée nationale a aussi repris plusieurs mesures de clarification ou de simplification

L'Assemblée nationale a également rejoint le Sénat sur l'essentiel des modifications techniques que la commission des finances avait portées à l'article 68 relatif à l'interdiction de l'octroi de garanties de l'État au commerce extérieur

nous ne pouvons que regretter, comme nous l'avons fait tout au long de la première partie, que le Gouvernement ait renoncé à redresser les comptes publics. J'avais expliqué, en première lecture,

tant en première qu'en seconde partie, l'Assemblée nationale ait rétabli, en nouvelle lecture, certaines dispositions auxquelles le Sénat s'était fortement opposé.

proposés par la commission des finances et adoptés par le Sénat à une très large majorité concernant le schéma de financement des collectivités territoriales. Monsieur le secrétaire d'État, je vous rappelle qu'Alain Richard, membre de La République En Marche,

une baisse du niveau des pensions et un changement de philosophie qui ouvrent la porte, à terme, qu'on le veuille ou non, à un système par capitalisation, provoquant l'inquiétude grandissante de nos concitoyens.

À rebours de ce que la rédaction de la motion laisse entendre, nous saluons les efforts accomplis en matière de maîtrise des comptes publics. Comme nous l'avons déjà dit ici même, nous aurions souhaité que ces efforts fussent plus ambitieux ; mais un principe de réalité s'impose.

Pourtant, les réserves ne manquent pas. Et pour cause : élus à la chambre des territoires, nous avons toujours à coeur de relayer et de faire valoir les revendications des collectivités territoriales et des acteurs du terrain. Cette année, ces revendications ont une pertinence toute particulière, puisque ce budget est d'abord celui de la fiscalité

L'Assemblée nationale aurait pu, sur ce point, se ranger à la sagesse du Sénat sans pour autant retarder la mise en oeuvre de la réforme ou en modifier profondément l'architecture. Même cas de figure concernant la rationalisation du dispositif de mécénat pour les grandes entreprises : si l'argument financier ne peut laisser insensible, une approche trop comptable risque, en l'occurrence, de priver les acteurs de terrain de financements vitaux pour le tissu associatif. Car rationaliser le dispositif de mécénat pour les versements importants, c'est tarir des ressources qui manquent déjà. L'Assemblée nationale a choisi d'ignorer les modifications que nous avions votées à la quasi-unanimité. C'est regrettable Cette mesure introduit de l'incertitude autour d'un dispositif qui brillait notamment par sa lisibilité et par sa stabilité, ce qui n'est pas si courant dans notre pays ; elle instaure en outre une forme de hiérarchisation des causes. Notre groupe a été force de propositions. Il a notamment cherché à encourager les collectivités à s'engager de façon volontaire dans la transition écologique. Ainsi notre proposition, largement partagée ici, visant à ouvrir le FCTVA à la location de véhicules électriques et hybrides constituait-elle une réponse pragmatique à un besoin exprimé par les élus locaux ; son adoption aurait fait avancer concrètement la transition écologique. Elle a connu le même sort que plusieurs de nos propositions ; nous le regrettons amèrement. De même, nous soutenions la position de sagesse arrêtée par la commission des finances concernant la taxe forfaitaire sur les CDD d'usage. Notre groupe en avait proposé la suppression pure et simple, mais le décalage dans le temps nous paraissait à la fois nécessaire et raisonnable. Nous regrettons que cette proposition n'ait pas été retenue. En définitive, le budget tel qu'il nous est présenté affiche affiche un recul du déficit nominal. Le volet des dépenses aurait pu, et aurait dû, compte tenu de la conjoncture favorable, être plus ambitieux en matière d'économies. Mais nous nous réjouissons que les budgets régaliens aient été sanctuarisés. Je pense notamment à la mission « Défense », dont j'ai eu l'honneur d'être l'un des rapporteurs.

le groupe Les Indépendants soutient une politique ambitieuse de réduction des dépenses publiques, tant que celle-ci ne se fait pas au détriment des fonctions régaliennes de l'État. De nombreuses améliorations peuvent encore être accomplies en matière de rationalisation de l'action publique, sans que cela nous pénalise collectivement face aux grands défis auxquels notre pays devra faire face. La parole est

le groupe Union Centriste votera dans sa grande majorité la question préalable. Très bien ! Nous remercions le rapporteur général d'avoir accepté d'amender la première version de son

Nous n'avons toujours pas les outils indispensables à une mesure efficace de l'impact budgétaire de nos propositions. La forteresse de Bercy est demeurée inviolable

Ce n'est pas dans de telles conditions que le Parlement peut accomplir sa mission pourtant fondatrice qu'est l'élaboration du budget de la Nation. Troisième frustration : des propositions de fond

inopportun. Je me permettrai donc de regretter la volonté de la majorité présidentielle et du Gouvernement de ne pas entendre la parole du Sénat et de mettre en oeuvre une démarche systématique de détricotage des travaux de la Haute Assemblée.

Concernant le fond, cependant, nous considérons qu'il ne nous appartient pas d'arbitrer entre un projet de loi de finances de droite et un projet de loi de finances de droite. Allons Les deux sont de droite

; engager une transition écologique réelle et non plus d'affichage ; encourager nos territoires. C'est à nos concitoyens, désormais, de se faire une opinion sur les orientations politiques retenues par le Gouvernement et par la majorité sénatoriale.

Cependant, mes chers collègues, plusieurs considérants énoncés par le rapporteur général nous conduiront à nous abstenir sur la motion tendant à opposer la question préalable. Si nous pouvons en effet vous rejoindre pour dénoncer la méthode de travail du Gouvernement, les constats politiques que nous formulons divergent assez largement. La parole

En effet, l'Assemblée nationale a achevé ses travaux tard la nuit dernière. Mes collègues du groupe du RDSE et moi-même comprenons cette situation, bien que cela limite, à nos yeux, les prérogatives du Sénat, dans le contexte social difficile que nous traversons en ce moment. Nous le répétons chaque année, les conditions d'examen du projet de loi de finances sont très particulières et ne sont pas toujours idéales. Des délais très contraints pour prendre connaissance du texte et pour proposer des amendements, avec l'obligation d'examiner l'ensemble en seulement vingt jours, nous conduisent bien souvent à survoler les différents sujets, qui sont pourtant nombreux et techniques. Acte très politique, le vote du budget traduit le soutien accordé ou non à la politique du Gouvernement. C'est pourquoi l'échec de la commission mixte paritaire faisait, comme chaque année, peu de doute. Avec près de 2 500 amendements déposés en première lecture, nous avons de nouveau battu un record. Je rappelle qu'il y avait eu 2 000 amendements l'an dernier, 1 400 amendements en 2017 et « seulement » 1 000 amendements en 2015. L'explication de Vincent Delahaye, qui

Comme je l'ai déjà souligné à l'issue de la première partie, je rappellerai de nouveau ici la place pivot de ce budget à la moitié du quinquennat. En première lecture, le Sénat avait reporté d'un an la réforme du financement des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale, lundi, a rétabli sa version, en adoptant une très longue série d'amendements. Elle a également supprimé les nombreuses niches fiscales introduites par la majorité sénatoriale, en particulier sur l'IFI (impôt sur la fortune immobilière) ou encore sur les droits de succession et les donations.

Je regrette, pour ma part, la suppression de dispositions adoptées sur l'initiative de membres de mon groupe tant sur la fiscalité du numérique qu'en ce qui concerne l'agriculture ou l'aménagement du territoire.

En ce qui concerne la fiscalité du numérique, comme je l'ai souligné, l'assujettissement des « pure players » du commerce en ligne à la taxe sur les surfaces commerciales répondait à une question d'équité fiscale, notamment par rapport aux acteurs traditionnels. Sur la fiscalité énergétique, nous avons soutenu avec succès des modes de chauffage renouvelables et l'usage de carburants alternatifs. La fiscalité environnementale ne doit pas s'opposer aux activités agricoles, elle doit au contraire être complémentaire nous l'avons montré dans des domaines cruciaux comme l'apiculture ou la protection des espaces forestiers. En matière d'aménagement du territoire, nous avons défendu, comme chaque année, la cause des territoires ruraux et enclavés, avec la préservation des petites lignes aériennes dans le cadre de la hausse de la taxe sur les billets d'avion, mais aussi les activités de montagne et la préservation des zones de revitalisation rurale.

comme celles des départements d'Île-de-France face aux atermoiements du financement du Grand Paris. Raté ! Nous en connaissions le résultat Mes chers collègues, gardons à l'esprit qu'il s'agit d'une loi de finances initiale. Si son examen prend beaucoup de temps et d'énergie, cela reste un budget prévisionnel. La « sincérisation » des lois de finances depuis 2017 est saluée par tous. Toutefois, il est impossible d'éviter un décalage entre la prévision et l'exécution, car les hypothèses macroéconomiques- croissance, inflation, etc. -sont, par définition, difficiles à anticiper. C'est pourquoi le projet de loi de règlement de l'été et les missions de contrôle budgétaires doivent être revalorisés. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le contexte européen. Aux élections générales du 12 décembre dernier, le peuple britannique semble avoir confirmé sa volonté de quitter l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Par ailleurs, la situation économique et politique d'autres voisins comme l'Italie reste préoccupante. Partout, les modèles politiques et sociaux sont remis en cause. Notre débat budgétaire en subit les conséquences. Ainsi, et il faut le déplorer, la gestion de la dette pèse inévitablement sur toutes nos politiques publiques. À ce propos, je mentionnerai le récent film de Costa-Gavras, qui met en scène les âpres négociations qui ont eu lieu il y a quelques années sur le programme d'aide au désendettement de la Grèce. Il montre combien les questions budgétaires et le bon fonctionnement de la démocratie sont intimement liés.

pour les acquisitions de terrains à bâtir destinés à des opérations de logement social. Ces deux modifications ont été finalement prises en compte et figurent dans le texte final. De même, en ce qui concerne l'encadrement de l'article 57 sur l'utilisation des réseaux sociaux par le fisc, tous nos apports ont été conservés. pour les foncières solidaires chargées d'un service d'intérêt économique général dans le domaine du logement

presse, les véhicules des collectivités territoriales ou la dotation destinée à compenser les frais d'assurance supportés par les communes de moins de 3 500 habitants

il paraissait impossible de trouver un accord global sur un texte qui comportait plus de 400 articles- un record sous la V République -, dont 238

Le Gouvernement a choisi de ne retenir aucun de nos amendements, ce que je regrette. Prenons le pari que les effets de bord seront considérables et que certaines dispositions reviendront dans le PLF de l'année prochaine, car vous nous avez d'ores et déjà annoncé une phase de révision, Je vous ai notamment entendu dire que toutes les questions relatives aux impacts sur le calcul des potentiels financiers et fiscaux seront à l'ordre du jour du CFL, qui se réunira au mois de janvier Il n'aurait pas été déshonorable d'accepter de reporter la mise en oeuvre de la réforme d'une année pour se donner le temps, tous ensemble, de faire des simulations et d'évaluer les conséquences sur chacune de nos collectivités.

par ailleurs la fiscalité écologique. Le PLF pour 2020 devait incarner l'orientation du Gouvernement vers un verdissement de sa politique.

Nous continuons de dénoncer cette fiscalité ; vous continuez de ne pas nous écouter. La majorité présidentielle a choisi de maintenir la suppression des comptes d'affectation spéciale, qui permettent pourtant une traçabilité de cette fiscalité : c'est une erreur. Pour incarner au plus près des territoires le tournant vert de votre politique, le Sénat, pour la quatrième année consécutive, a voté à l'unanimité une affectation partielle des recettes de la TICPE aux régions et aux EPCI. À travers les plans territoriaux et les schémas régionaux, ces acteurs mènent des actions concrètes et visibles des citoyens. L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Mesure au coût anecdotique- 300 000 euros -, mais forte en symboles, le bénéfice du FCTVA pour la location longue durée d'un véhicule à faibles émissions par les collectivités locales a également été rejeté par les députés. Le Sénat, à l'unanimité, l'avait pourtant voté. Je m'interroge sur les capacités des collectivités à atteindre les objectifs qui leur ont été fixés dans la loi d'orientation des mobilités. Autre exemple : le domaine de la culture, qui a déjà été largement évoqué par le rapporteur général et lors des questions d'actualité au Gouvernement. Notre groupe croit à la nécessité de préserver le patrimoine historique de notre pays. Après la baisse des crédits du patrimoine dans le projet de loi de finances rectificative, nous nous demandons si ce souci est partagé par le gouvernement actuel. Il est vrai que le Président de la République, alors en campagne, avait expliqué qu'il n'y a pas de « culture française ». Chacun connaît les difficultés pour les particuliers d'entretenir des demeures historiques, qui sont des gouffres financiers. L'impôt sur la fortune immobilière les pénalise fortement alors qu'ils ne retirent aucun bénéfice de leur bien ouvert au public, les recettes étant réinjectées pour l'entretien et la rénovation. Cela fait par ailleurs travailler les entreprises et préserve un savoir-faire artisanal français unique. Le Sénat avait proposé d'exonérer d'IFI à hauteur de 75 % les monuments historiques ou classés en zone rurale, ouverts au public, avec un engagement de conservation. Quelle est la justification du rejet de cette mesure ? Quelle raison justifie également la suppression de l'exonération de taxation pour le loto du patrimoine ou encore la réforme du mécénat d'entreprise, rétablie à l'Assemblée nationale, qui va faire économiser environ 20 millions d'euros sur le mécénat patrimonial ? Le dernier exemple, enfin, est la lutte contre la fraude. Comme l'an passé, nous constatons avec regret que vous ne voulez toujours pas reprendre notre proposition de lutte contre la fraude aux dividendes : vous la jugez mal calibrée. Pourtant, nous reprenons le dispositif mis en place par les Allemands, dispositif qui va leur rapporter un montant considérable. L'outil que vous avez mis en oeuvre en juillet, figurant à l'article 119 A du code général des impôts, est calibré bien au-dessous de ce que nous proposons. L'Autorité des marchés financiers avait estimé que notre proposition pourrait rapporter entre 1 milliard et 3 milliards d'euros aux caisses de l'État. Peut-être aurons-nous raison dans un an ? Comme toujours ! Vous aviez rejeté les propositions de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude à la TVA. Je constate qu'elles ont fini par être reprises dans le présent budget. Nous le voyons à travers ces exemples, le fossé qui sépare la majorité sénatoriale de la majorité présidentielle est bien trop grand pour qu'un quelconque accord puisse être espéré. Nous le regrettons, car notre démarche au Sénat est celle d'une opposition constructive. Avant de conclure, je ne peux manquer de relever trois faits surprenants qui concernent directement mon département. Ah ! L'Assemblée nationale a rétabli la surtaxe sur les bureaux dans une zone dite « premium ». C'est une augmentation de 32 % en deux ans d'un impôt de production. Quelle logique avec la politique globale du Gouvernement en matière d'économie ! Le Sénat, à l'unanimité, a supprimé le prélèvement d'une fraction des droits de mutation des départements franciliens pour financer la part État du contrat de plan État-région porté par la Société du Grand Paris. Les départements vont venir se substituer à l'État alors même qu'ils ne sont pas compétents pour la politique des transports depuis la loi NOTRe, exception faite du transport des élèves souffrant d'un handicap. On marche sur la tête Enfin, les communes franciliennes contributrices au Fonds de solidarité de la région Île-de-France paieront plus que leur contribution naturelle pour compenser une mesure de plafonnement qui ne s'applique qu'à la Ville de Paris. Concernant cette augmentation du fonds, je relève qu'elle a une nouvelle fois été votée sans aucune étude d'impact et sans véritable argument la justifiant. C'est mon troisième PLF, et j'ai l'impression que chaque année nous rejouons exactement la même pièce avec une certaine frustration, comme l'a relevé mon collègue Delahaye. Le Sénat n'est pas plus écouté qu'avant, malgré les précédents fâcheux pour le Gouvernement et le niveau de tension rarement atteint dans notre pays. Vous vous privez du corps intermédiaire des parlementaires, avec un Sénat ostracisé et une Assemblée nationale qui s'apparente plutôt à une simple chambre d'enregistrement. Dans ces conditions, il est inutile de refaire le débat et de réexaminer le budget : les mêmes causes auront en effet les mêmes conséquences. C'est pourquoi le groupe Les Républicains approuvera la position de la commission des finances et votera la motion tendant

du Sénat. Monsieur le rapporteur général, à vos yeux, l'Assemblée nationale et le Gouvernement n'ont pas retenu suffisamment de dispositions adoptées par le Sénat. Le sénateur Bargeton a eu raison de souligner, comme j'avais commencé à le faire,

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 27 novembre dernier pour examiner les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille est parvenue à un accord. Cet accord a été rendu possible grâce à l'engagement et au sens des responsabilités de l'ensemble des députés et des sénateurs qui y siégeaient. Il n'était pas envisageable, à nos yeux, de terminer sur un constat d'échec, qui aurait retardé l'entrée en vigueur de plusieurs mesures attendues par nos concitoyens- je pense notamment à la réforme de l'ordonnance de protection et à l'entrée en vigueur du bracelet anti-rapprochement. Chacun a fait des concessions en gardant à l'esprit l'objectif qui nous rassemble tous : mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. Je ne m'attarderai pas sur les dispositions pénales dans la mesure où le texte issu des travaux de la CMP retient, pour l'essentiel, les rédactions que le Sénat avait adoptées. Nos discussions ont davantage porté sur le volet civil. La commission mixte paritaire est revenue sur des dispositions que le Sénat avait adoptées, contre l'avis de la commission, concernant le dépôt de plainte et les modalités d'assignation dans le cadre d'une ordonnance de protection. Il nous a semblé que ces dispositions pourraient se révéler contre-productives en introduisant des éléments de rigidité dans ces procédures. a également prévu que la possibilité donnée au juge aux affaires familiales d'ordonner le recours au bracelet anti-rapprochement serait évaluée au bout de trois ans, mais sans en faire un dispositif expérimental, ce qui nous a semblé constituer un compromis acceptable. La CMP n'a pas non plus retenu les articles additionnels que le Sénat avait introduits au sujet de l'indignité successorale. Nous avions voulu, en insérant ces articles, envoyer un message politique clair : la solidarité qui existe normalement entre époux n'a plus lieu d'être lorsqu'un conjoint commet des violences sur l'autre membre du couple. Nos collègues députés ont estimé que la réflexion n'avait pas suffisamment mûri sur ce point, qui pourra cependant être réexaminé dans le cadre de la prochaine proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, déposée par les députés Bérengère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha. La CMP a en revanche retenu l'article additionnel que nous avions adopté tendant à priver le conjoint violent du bénéfice de la pension de réversion. Elle en a même élargi le champ d'application, afin qu'il ne concerne pas seulement les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale. L'essentiel de nos débats a porté sur la question du retrait de l'autorité parentale, sur laquelle je voudrais m'arrêter quelques instants. Avec notre collègue Aurélien Pradié, rapporteur de l'Assemblée nationale, j'ai proposé d'inscrire dans le texte un article reprenant l'une des principales propositions issues du Grenelle contre les violences conjugales. Trop souvent, lorsqu'une femme quitte le domicile pour échapper à la violence, son mari parvient à la retrouver parce qu'il a conservé l'autorité parentale et qu'il sait donc où sont scolarisés les enfants. Pour la sécurité des femmes, il est donc important de prévoir une suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale, dans l'attente de la décision d'un juge. Absolument ! Sur le fond, cette mesure a suscité un large accord parmi nos collègues députés et sénateurs. Certains auraient préféré disposer de plus de temps pour en étudier les aspects techniques, mais nous avons estimé qu'il était urgent de légiférer sur ce sujet, dans l'intérêt des femmes victimes de violences conjugales et surtout de leurs enfants. Je vous présenterai tout à l'heure un amendement, qui a donné lieu à des échanges avec l'Assemblée nationale et le Gouvernement, afin d'en peaufiner la rédaction et de corriger les quelques imperfections qui subsistent. En ce qui concerne, enfin, le volet du texte destiné à faciliter le relogement des victimes, la commission mixte paritaire a procédé à des retouches mineures, destinées à mieux associer les parlementaires au bon déroulement des expérimentations proposées. proposées. Mes chers collègues, je me réjouis que le travail réalisé en commun sur ce dossier des violences conjugales ait abouti, en seulement quelques mois, à l'adoption d'un ensemble de mesures qui vont apporter des réponses concrètes à la détresse de trop nombreuses victimes. Je ne prétends pas que ce texte est la solution à tous les problèmes que celles-ci rencontrent, et il nous reste évidemment encore beaucoup à faire. D'autres mesures législatives sont en cours de préparation, dont nous débattrons l'année prochaine, avec le même esprit d'ouverture. Il faut en convenir, de nombreuses actions à mettre en oeuvre ne relèvent pas de la compétence du législateur. Je ne doute pas que le Gouvernement veillera à lancer dans les meilleurs délais les marchés publics nécessaires au déploiement du bracelet anti-rapprochement. Il est essentiel, en parallèle, de travailler sur la qualité de l'accueil des victimes dans les postes de police et de gendarmerie afin que leur parole soit convenablement entendue. Par ailleurs, les associations qui accompagnent les victimes et font de la prévention doivent être soutenues, ce qui suppose de mobiliser les moyens budgétaires adéquats. Au-delà, c'est tout un travail d'éducation et de sensibilisation qui doit être mené, dans la durée, afin que notre société ne tolère plus qu'un homme- c'est le cas le plus fréquent -lève la main sur sa compagne ni qu'il la rabaisse ou qu'il l'humilie, car les violences psychologiques constituent aussi un fléau que nous devons combattre. Nous devons faire passer l'idée auprès de nos concitoyens que la violence est non pas une manifestation de force, mais au contraire une marque de faiblesse et un échec de la communication, de la parole. Sur tous ces chantiers, le Gouvernement sait qu'il pourra compter sur le soutien vigilant

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure- chère Marie Mercier -, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs,

quelle que soit notre appartenance politique. C'est dans cet esprit que le Premier ministre a ouvert, le 3 septembre dernier, le Grenelle contre les violences conjugales et que le Parlement a adopté, en commission mixte paritaire, la proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise. Dans la lutte contre les violences conjugales, la justice occupe évidemment une place centrale. Je mène à ce titre, depuis plusieurs mois, une action volontariste, fondée sur un plan très structuré. La circulaire du 9 mai dernier, que j'ai adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, érige en priorité de politique pénale la lutte contre les violences faites aux femmes et incite les parquets à utiliser pleinement l'arsenal législatif dont ils disposent, comme les téléphones grave danger ou l'ordonnance de protection. que le recours à cette ordonnance de protection soit facilité et devienne une pratique régulière, presque un réflexe. Mes services ont d'ailleurs récemment analysé

La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui vise, d'une part, à renforcer l'ordonnance de protection et, d'autre part, à généraliser l'utilisation du bracelet anti-rapprochement (BAR). Je partage cette double volonté, puisqu'elle correspond aux aux deux axes majeurs sur lesquels travaille le ministère de la justice depuis plusieurs mois. Concernant l'ordonnance de protection, afin d'accroître le recours à ce dispositif très protecteur qui permet au juge aux affaires familiales d'organiser la séparation du couple dans un contexte de violences, il est prévu que la victime puisse obtenir, par une même décision de justice, des mesures à la fois civiles et pénales mesures civiles concernant l'organisation de la vie familiale, notamment les droits de visite et d'hébergement, la pension alimentaire ou encore l'attribution du logement du couple ; mesures pénales, telles que l'interdiction d'entrer en contact et l'interdiction de port d'arme. Le texte qui vous est soumis prévoit que le juge aux affaires familiales devra désormais statuer dans un délai de six jours à compter de la date de fixation de l'audience. Afin que ce délai soit effectif, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'ordonnance de protection devront être adaptées. Mes services y travaillent déjà. La proposition de loi apporte également des précisions indispensables. J'en cite quelques-unes à titre d'exemple : une plainte pénale n'est pas nécessaire pour demander une ordonnance de protection les auditions peuvent se tenir séparément si la partie demanderesse le souhaite ; l'ordonnance de protection peut être délivrée aux couples qui ne cohabitent pas et n'ont jamais cohabité. Ces précisions et d'autres encore ont une vertu pédagogique et nous permettent de répondre aux recommandations formulées par le Grevio, le groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dans son rapport d'évaluation sur la France, publié le 19 novembre dernier. Notons que le Grevio « salue la grande détermination dont les autorités françaises font preuve pour inscrire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes parmi leurs priorités politiques. » Il souligne également que l'adhésion des autorités à cette cause a été renforcée d'initiatives récentes, telles que le premier Grenelle contre les violences conjugales lancé par le Gouvernement le 3 septembre 2019. S'agissant du bracelet anti-rapprochement, il pourra être imposé aux auteurs de violences conjugales à titre de peine, mais aussi avant tout jugement pénal dans le cadre d'un contrôle judiciaire

Je crois profondément que ce nouveau dispositif, dédié à la seule protection des victimes, pourra éviter un nombre important de féminicides, comme cela a été le cas en Espagne. La proposition de loi initiale a été enrichie par de nouvelles dispositions concernant l'autorité parentale. Au moment du passage de la présente proposition de loi dans cet hémicycle, ces dispositions faisaient encore l'objet de concertations. La commission mixte paritaire a, par la suite, fait le choix de les inclure dans le texte que nous examinons aujourd'hui, sans attendre un nouveau véhicule législatif. Figurent ainsi deux mesures nouvelles. La première- Mme la rapporteure l'a précisé -ouvre au juge pénal la possibilité de statuer sur le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement. Cette disposition, qui offre plus de souplesse au juge, est de nature à lui permettre de mettre en oeuvre une solution plus adaptée à la situation familiale lorsque le retrait de l'autorité parentale paraît trop radical. La seconde mesure crée une suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, et ce dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales. Mme la rapporteure vous proposera tout à l'heure un amendement visant à préciser la rédaction de cet article. Le Gouvernement y sera favorable. La lutte contre les violences au sein du couple va se poursuivre. Il est désormais temps de tirer les enseignements des travaux menés dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, ainsi que de ceux menés par les députés du groupe La République En Marche à l'issue de leurs journées de travail en région. Ces réflexions ont conduit à formuler de nombreuses propositions. Plusieurs d'entre elles sont convergentes avec les réflexions et travaux menés dans le cadre du groupe de travail « Justice » que j'ai installé à la Chancellerie à la suite du lancement du Grenelle. Ce groupe de travail continuera d'ailleurs ses travaux afin de suivre l'avancée des actions qui ont été annoncées. Il s'agit en effet d'inscrire notre action dans la durée, au-delà même de la séquence du Grenelle. Parmi les nombreuses propositions formulées par les députés, certaines exigeaient des modifications de nature législative. Elles trouvent leur expression dans la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, déposée le 3 décembre dernier par les députés de La République En Marche. Cette proposition de loi sera discutée dans les semaines à venir et connaîtra également-

pénale ainsi qu'à assurer l'organisation de la vie de famille et la protection effective des victimes de violences familiales, qu'il s'agisse des parents ou des enfants. proposition de loi tend à inscrire dans la loi que les enfants ne seront plus tenus d'aucune obligation alimentaire à l'égard du parent qui aura tué l'autre parent, tué l'autre parent, à proscrire toute médiation, tant civile que pénale, en cas de violence et en cas d'emprise, ce qui répond à une demande très forte des associations, et à permettre et à permettre aux médecins de révéler plus facilement les faits de violences conjugales à la justice, même en l'absence d'accord de la victime, dans certaines circonstances particulières rigoureusement encadrées. encadrées. Elle prévoit par ailleurs d'étendre l'incrimination de certains comportements et de favoriser leur répression, notamment en sanctionnant plus sévèrement le harcèlement au sein du couple qui aura conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire et en pénalisant plus largement les comportements d'espionnage. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je tiens, comme l'a fait Mme la rapporteure, dont je salue le travail, à vous assurer de l'engagement absolu du ministère de la justice sur ce sujet, et du mien en particulier. Nous continuerons, avec l'aide de tous, non seulement des magistrats et des forces de l'ordre, mais aussi des avocats, des réseaux associatifs et de l'ensemble de la société civile, à lutter contre des actes qui, en meurtrissant chaque jour des femmes, heurtent la société tout entière. J'en suis absolument certaine,

parce qu'elle vise à prévenir ces violences et à les punir, la proposition de loi que nous adopterons aujourd'hui revêt une importance capitale. Une femme sur trois dans le monde est exposée à la violence au cours de sa vie. Le plus souvent, cette violence s'exerce au sein même du couple. Parce qu'elles représentent une altérité et que leur liberté ne coïncide pas toujours avec celle des hommes, les femmes sont souvent victimes d'un engrenage de violence, qui commence par des mots, des menaces et finit par des coups. Parfois, mais toujours trop souvent, ces coups sont mortels. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 38 % des meurtres de femme sont le fait de leur conjoint ou ex- conjoint. Ces violences domestiques sont les derniers vestiges de mentalités arriérées, d'un sexisme primaire, d'une relation d'oppression insupportable. L'égalité entre les femmes et les hommes devrait être non pas une question, mais une évidence. Pour reprendre les mots de Simone Veil, il s'agit non pas d'effacer les différences, mais de les prendre en compte. En parallèle des travaux parlementaires, le Gouvernement a engagé un Grenelle contre les violences conjugales en septembre dernier pour apporter le plus rapidement possible des solutions opérantes et efficaces pour protéger les victimes. Dix mesures d'urgence ont été annoncées, aux premiers rangs desquelles figurent la création de 1 000 nouvelles places d'hébergement, un audit général des commissariats et des gendarmeries et la possibilité de déposer plainte à l'hôpital. D'autres mesures suivront, début 2020, pour inscrire dans la loi les propositions issues de la concertation nationale. La proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille sein de la famille est l'initiative du député Aurélien Pradié, dont nous saluons ici le travail. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord le 27 novembre dernier, preuve que cette question rassemble toutes les sensibilités politiques- c'est heureux ! -et que chacun d'entre nous est prêt à s'engager pour protéger davantage les femmes victimes de ces violences. Les deux principales mesures dont bénéficieront directement les victimes sont la généralisation du bracelet anti-rapprochement et la réduction du délai maximal de délivrance de l'ordonnance de protection à six jours au lieu de quarante-deux jours. Le dépôt de plainte ne sera plus nécessaire à sa délivrance. Au cours de son examen, notre assemblée a largement contribué à enrichir le texte, avec des dispositions importantes. Je citerai notamment la sensibilisation des jeunes à la lutte contre les violences conjugales lors de la journée défense et citoyenneté et la succession du conjoint condamné pour des faits de violence envers le défunt. La commission mixte paritaire a souhaité supprimer cette dernière mesure, et nous le regrettons. Nous saluons la bienveillance de la commission à l'égard de la demande de rapport sur les conséquences du maintien de l'autorité parentale de l'auteur de violence et la possibilité de sa suspension. Nous invitons le Gouvernement à aller plus loin que la production d'études et de rapports qui, trop souvent, ne font qu'alourdir les étagères des bureaux ministériels. La commission mixte paritaire a conforté l'article 2 relatif à l'ordonnance de protection, tout en limitant à l'article 2 l'utilisation d'un bracelet anti-rapprochement à une durée initiale de trois ans, renouvelable selon l'appréciation du juge. Il s'agit là du coeur de la proposition de loi. Proposé par le Gouvernement, l'article 2 inscrit au Fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes les personnes visées par une ordonnance de protection. Nous sommes bien sûr favorables à ce dispositif de bon sens. En juillet dernier, 150 sénateurs alertaient le Gouvernement et l'opinion publique avec la publication d'une tribune appelant à une généralisation des bracelets électroniques pour prévenir les féminicides. Quelques mois plus tard, cette initiative menée par Annick Billon et la délégation aux droits des femmes a trouvé un écho à travers cette proposition de loi issue de l'Assemblée nationale. Le groupe Les Indépendants - République et territoires renouvelle son soutien : nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille traduit une véritable prise de conscience de l'effroyable réalité que représentent les violences intrafamiliales. À l'occasion de l'examen du texte en première lecture, le 27 novembre dernier, nous étions nombreux à rappeler combien de femmes avaient succombé sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année 2019. Elles sont aujourd'hui 142 selon le collectif Féminicides. Il est temps que ce décompte macabre s'achève et que nous nous dotions des moyens judiciaires, humains et financiers suffisants pour que ce fléau cesse. Aussi, je me réjouis de l'aboutissement de cette commission mixte paritaire, qui traduit notre volonté, au-delà des clivages politiques, de trouver des solutions afin de mieux lutter contre ce fléau. C'est aussi grâce à J'en profite pour remercier le président Philippe Bas et la rapporteure Marie Mercier de leur investissement, ... Surtout Marie Mercier ! ... qui a permis d'aboutir à une CMP conclusive. Les violences au sein de la famille sont souvent difficiles à caractériser et à dénoncer, car elles pâtissent encore de nombreux stéréotypes. Pour exemple, les mots « crime passionnel » persistent encore dans certains esprits. Souvent minorées et considérées comme relevant de la sphère intime, ces violences relèvent avant tout d'un caractère systémique et nécessitent d'interroger de façon plus générale les rapports de domination qui animent notre société. Nous avons, nous, législateurs, une responsabilité forte et une capacité d'action pour faire baisser ces violences. Cette CMP est fondamentale dans la mesure où elle propose de compléter notre arsenal juridique par des avancées concrètes en matière de protection des victimes de violences conjugales. La mise en place du bracelet électronique anti-rapprochement au début de l'année prochaine, les aides au logement, les modalités de recours au téléphone grave danger, la facilitation de la délivrance de l'ordonnance de protection constituent autant de mesures concrètes et attendues qui amélioreront de manière significative la protection des femmes. Je me félicite tout particulièrement que la question de l'autorité parentale, que j'avais portée avec la délégation aux droits des femmes, ait été reprise à la faveur de cette CMP, même si cette disposition ne va pas assez loin à mon sens : le caractère provisoire de la suspension de l'autorité parentale, d'une durée de six mois, en limite notamment sa portée. Les nombreux travaux de la délégation ont montré que, bien souvent, l'existence d'enfants permet l'exercice d'un chantage visant à poursuivre le harcèlement ou les violences sur l'ex-conjointe ; nous sommes convaincus qu'un mari violent ne saurait être un bon père. En effet, sans l'organisation adaptée des modalités d'exercice de l'autorité parentale, les mesures de protection de la femme victime de violences seront mises en échec et les enfants ne seront pas protégés. Une prise en compte élargie des violences conjugales est indispensable pour assurer une protection effective de la mère et de l'enfant. Dès lors, la suspension de plein droit de l'autorité parentale ne saurait se cantonner

dispenser les enfants de l'obligation d'aliment en cas de retrait total de l'autorité parentale et d'exclure cette obligation en cas de condamnation pour le meurtre ou l'assassinat de l'autre parent. J'ai regretté que cette proposition, pourtant consensuelle, ait été rejetée par le Gouvernement comment accepter qu'un enfant conserve une obligation d'aliment vis-à-vis de son parent auteur d'un assassinat sur son autre parent ? que vous avez rejetée, figure pourtant parmi les annonces du Gouvernement dans le cadre du Grenelle. Elle devrait donc trouver une transcription législative dans un prochain texte. Sans vouloir faire il eût été plus opportun de l'intégrer dans cette proposition de loi ; cela nous aurait fait gagner du temps, que nous savons précieux. Je souhaite terminer en évoquant une question fondamentale : la question financière. Si ce texte constitue une avancée indéniable, ses dispositions ne sauraient se concrétiser sans des moyens massifs. Je n'ai eu de cesse, au cours de mon mandat de présidente, que de déplorer le hiatus existant entre les ambitions affichées par le Gouvernement, dans le cadre de la « grande cause du quinquennat », et la réalité des moyens qui y sont consacrés.

Trop de familles se trouvent démunies face à la procédure judiciaire et aux frais de justice importants que celle-ci induit. La responsabilité qui nous incombe est forte, tout comme l'attente de notre société. Soyons à la hauteur des enjeux, soyons au rendez-vous ! Cette proposition de loi d'Aurélien Pradié, point de départ d'un combat que nous savons long, va dans le bon sens. C'est pourquoi le groupe Union Centriste, souhaitant encourager le travail accompli, votera ce texte.

à rester sous l'autorité parentale d'un père violent. Un père violent qui attaque la mère, qui s'en prend à elle, qui la brutalise, ne peut pas

une femme faisant l'objet d'une ordonnance de protection, mais à laquelle le juge n'aura pas attribué l'autorité parentale exclusive, sera exposée au risque que son conjoint violent la retrouve,

À l'heure où un 145 féminicide a été commis cette année, nous devons mettre tous les moyens de notre côté pour lutter contre la banalisation des violences faites aux femmes, mais aussi pour instaurer un régime plus protecteur des victimes, trop souvent laissées à l'abandon.

À ce titre, je salue les travaux menés par les commissions des lois des deux assemblées, qui ont permis d'aboutir à une CMP conclusive. Les apports du Sénat, visant à renforcer les garanties procédurales, ont été reconnus à leur juste valeur, et nous avons de quoi nous en satisfaire. Je veux citer l'article 2 , qui prévoit l'inscription des personnes auteurs de violences conjugales au Fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Cette disposition constitue, selon moi, une véritable avancée ; combien de fois un fusil de chasse s'est-il transformé en une pièce à conviction lors d'un féminicide ? Je note également l'exclusion de la succession du conjoint condamné pour des faits de violence envers le défunt ou encore l'exclusion du bénéfice de la pension de réversion, en cas de divorce,

Qu'une mesure si coercitive puisse être prise par un juge civil, sans la moindre condamnation, nous semble incompatible avec les fondements de notre droit pénal. Le risque est effectivement que l'ordonnance de protection se substitue au jugement pénal ; nous y sommes défavorables. Ma collègue l'avait déjà souligné, dans un contexte où seulement une demande d'ordonnance de protection sur deux aboutit, nous prônons plutôt la meilleure prise en compte des signaux dits

Ces mesures sont motivées par l'intérêt supérieur de l'enfant, qui ne doit pas, à notre sens, être confronté à des individus violents. Je ne vous apprendrai pas qu'un enfant ayant été confronté tôt à la violence a de très grandes chances de reproduire ce type de comportements. La solution est donc claire : si l'on souhaite enrayer la spirale de la violence, il faut séparer les enfants des parents violents. Conscients de l'urgence à apporter des solutions aux trop nombreuses victimes de violences et satisfaits de l'équilibre général trouvé au travers de ce texte, les élus du groupe du RDSE approuveront les conclusions de la CMP. Je veux remercier

dispositif, la victime de violences conjugales peut obtenir, au travers d'une même décision de justice, des mesures tout à la fois civiles et pénales. et pénales. Les mesures civiles concernent l'organisation de la vie familiale, avec, au premier chef, les droits de visite et d'hébergement, la pension alimentaire ou encore l'attribution du logement du couple. couple. Les mesures pénales sont relatives à l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et à l'interdiction, pour le conjoint violent, de port d'arme. second lieu, ce texte a été conçu pour sauver des vies, en généralisant l'utilisation du bracelet anti-rapprochement. Trop souvent, l'actualité s'est fait l'écho

Ainsi, le bracelet pourra être imposé aux auteurs de violences conjugales à titre de peine, mais aussi avant tout jugement pénal dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou, en dehors de toute plainte, dans le cadre civil d'une procédure d'ordonnance de protection. Nous approuvons, sans aucune réserve, l'ensemble de ces mesures. Néanmoins, une priorité absolue demeure : faire reculer les violences.

La réduction du délai de délivrance de l'ordonnance de protection est l'un des leviers d'action absolument nécessaires. Pour que cet objectif législatif soit entièrement effectif, il faudra non seulement ajuster en conséquence les dispositions du code de procédure civile relatives à l'ordonnance de protection, mais également poursuivre la revalorisation budgétaire de nos structures judiciaires, sans lesquelles notre opiniâtreté pourrait se dissoudre en voeux pieux. veux maintenant dire quelques mots sur l'heureuse issue des mesures relatives à l'autorité parentale. Nous avions déposé, en séance, un amendement ayant pour objet de suspendre de plein droit l'autorité parentale lorsque l'un des deux parents est décédé des suites d'un homicide volontaire et dont les faits font l'objet d'une enquête pénale mettant en cause l'autre parent, ou d'une information judiciaire ouverte à l'encontre de celui-ci. Pour assortir ce dispositif d'un brevet de respectabilité constitutionnelle, nous avions laissé toute liberté d'appréciation à la juridiction compétente, laquelle pouvait, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total, notamment lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le commandait.

une disposition analogue, qui prévoit la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, et ce dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales. Juridiquement, vous avez décidé d'ajuster le droit aux dimensions du réel, et le réel, en tout état de cause, ce sont les victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, le droit leur répond, la raison a prévalu. Nous ne pouvons que nous en féliciter,

une disposition qui n'avait, finalement, pas été adoptée par le Sénat et qui n'avait même pas été débattue par l'Assemblée nationale. Sans doute, nous aurions pu faire l'économie d'un désaccord de procédure qui nous a occupés,

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous arrivons au terme de cette navette parlementaire, et, je dois le dire, nous ressentons quelque frustration liée à la façon dont se sont déroulés les débats.

sous les yeux de leurs enfants. Si la question du féminicide, des violences contre les femmes et des agressions sexistes, notamment au sein de la famille, a pu devenir un véritable enjeu de société cette année, c'est grâce aux nombreuses mobilisations des femmes et des associations féministes. Cette loi en est aussi la conséquence, et c'est une bonne chose. Je veux revenir sur les principaux articles du texte. Nous saluons le fait que, en CMP, la discussion sur l'autorité parentale ait évolué et que nous passions ainsi d'un simple rapport sur le sujet à une suspension en cas de crime commis sur l'autre parent.

377 du code civil, qui traite de la délégation de l'autorité parentale, nous paraissait totalement inapproprié. Nous nous réjouissons vraiment de l'apport de l'amendement de notre rapporteure, Marie Mercier,

Nous l'avons dit et nous le répétons, l'hébergement d'urgence pour les personnes victimes de violences doit être la priorité, cela doit concentrer tous nos efforts. Au-delà de l'hébergement d'urgence, nous saluons l'effort accompli pour permettre aux femmes victimes d'accéder à un logement pérenne, avec un accompagnement financier.

Quant au bracelet anti-rapprochement, c'est un dispositif qui doit être utilisé avec prudence et discernement. S'il constitue un véritable outil dissuasif, reste en suspens la question de la distance requise pour tenir le conjoint violent éloigné, distance laissée à la discrétion du juge. Ce n'est pas une question anecdotique ; être éloigné de deux ou de vingt kilomètres n'aura clairement clairement pas le même effet anxiogène sur la victime, qui a bel et bien besoin d'un environnement sécurisant. De plus, lors du colloque que j'ai organisé salle Médicis le 22 novembre dernier, intitulé « Du sexisme ordinaire aux féminicides plusieurs intervenants, dont le magistrat Édouard Durand, nous ont alertés sur la difficulté pour les personnes victimes de violences- femmes et enfants -à rompre le lien avec leur agresseur. Cette emprise les place dans une grande dépendance, dont elles ont du mal à se défaire. Le bracelet électronique serait alors un obstacle supplémentaire au fait, pour la victime, de se défaire du lien. Ne serait-il pas plus efficace de développer le nombre de téléphones grave danger, qui ont fait la preuve de leur utilité ? Enfin- c'est le plus inquiétant, madame la garde des sceaux -, depuis la fin du Grenelle, nous avons discuté du projet de loi de finances pour 2020 ; ces véritables travaux pratiques ont été marqués par l'absence de garantie budgétaire pour le financement des places d'hébergement d'urgence, du logement temporaire et des bracelets anti-rapprochement, dont il est question dans cette proposition de loi. Je vous le demande donc : pouvez-vous nous rassurer sur les moyens

Le phénomène des violences conjugales, particulièrement médiatisé au cours des derniers mois, n'est pas récent. Rappelons-nous cette atroce banalité, si bien décrite par Zola, à la fin du XIX siècle, dans son célèbre roman. Déjà, à l'époque, le romancier s'interrogeait sur la racine de ce mal, qui poussait certains de ses personnages à commettre, parfois, l'irréparable. Cette terrible réalité nous oblige, et je me réjouis du caractère conclusif de cette commission mixte paritaire. Je m'en réjouis d'autant plus que plusieurs apports du Sénat ont prospéré au sein du texte adopté par cette commission. Ainsi en est-il de la possibilité, pour le juge aux affaires familiales, de délivrer une ordonnance de protection à tous les couples, donc même à ceux qui auraient mis un terme à leur vie commune ou qui n'auraient jamais fait le choix de cohabiter. Cette disposition simple me paraît néanmoins essentielle, puisqu'elle permettra, je le crois, de protéger davantage de femmes victimes de violences. L'article 2 , résultant également des travaux de notre commission des lois et qui est demeuré dans le texte issu de la commission mixte paritaire, constitue aussi une avancée souhaitable. En effet, il inscrit dans la loi l'interdiction, pour une personne condamnée pour des faits de violences conjugales, de bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de son ex-conjoint victime de ces violences. En outre, la position commune trouvée avec nos collègues députés, qui étend le bénéfice de cette disposition au-delà des seuls salariés du secteur privé, me paraît encore plus pertinente. Avec un peu de recul, une telle mesure nous semble presque relever du bon sens. Je ne peux, bien sûr, faire l'impasse sur la mesure phare de cette proposition de loi de notre collègue député Pradié : le bracelet anti-rapprochement. Une position de compromis a ainsi été trouvée entre les deux chambres, puisque l'efficacité du dispositif sera évaluée dans les trois ans qui suivront la promulgation de la loi. Il nous semblait souhaitable de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à un dispositif aussi inédit que celui-ci, en matière civile. Il conviendra notamment d'apprécier de quelle manière les juges aux affaires familiales s'en seront saisis et si ce bracelet aura effectivement permis de répondre à des situations de danger. Il est heureux que les députés aient pris en considération la volonté de prudence du Sénat en la matière. Malgré l'accord trouvé sur le texte en commission, deux problématiques ont toutefois provoqué des débats mouvementés. Je souhaite les évoquer brièvement.

L'absence de véritable navette parlementaire, du fait de l'engagement, par le Gouvernement, de la procédure accélérée sur ce texte, n'a en effet pas permis aux députés d'examiner cette question. Cela est regrettable. l'autre difficulté que nous avons rencontrée portait sur la question de la suspension de l'autorité parentale d'un parent auteur de violences au sein de la famille, question encore plus sensible que la précédente, dans la mesure où elle risque de se poser au juge de manière beaucoup plus récurrente. Je pense que la solution à laquelle nous sommes parvenus, après de longues discussions en CMP, est raisonnable. En permettant au juge de suspendre l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, nous avons adopté une disposition qui envisage les cas les plus graves. sera toutefois nécessaire de légiférer plus avant sur ce sujet. L'objet spécifique de cette proposition de loi ne permettait peut-être pas de traiter la question en toute sérénité. Sans doute aussi les députés ont-ils préféré attendre le texte porté par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Pour conclure, je tiens à remercier notre rapporteur, Marie Mercier, de la qualité de son travail. Elle a su faire preuve de beaucoup d'humanisme à propos d'un sujet particulièrement sensible. Bien évidemment, le groupe Les Républicains est satisfait du caractère conclusif de la commission mixte paritaire et votera cette proposition de loi. La discussion générale est

examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement. Je donne lecture du texte élaboré par la commission

relatif au retrait de l'autorité parentale, sans modifier l'équilibre du texte approuvé par la commission mixte paritaire. Le paragraphe I tend à préciser que, si l'un des parents a commis un crime sur la personne de l'autre parent, peut être saisi pour décider de déléguer l'exercice de l'autorité parentale seulement lorsque le parent victime a perdu la vie. Dans le cas contraire, il revient naturellement au parent victime de continuer à assurer l'exercice de l'autorité parentale, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une délégation. du paragraphe II a pour objet de préciser que la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale prévue en cas de condamnation s'applique y compris lorsque la condamnation n'est pas définitive. Sinon, il suffirait d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation pour que cette disposition soit privée d'effet.

relatif à la délégation de l'autorité parentale. En fonction des circonstances de l'espèce, d'autres procédures prévues par le code civil peuvent en effet apparaître plus appropriées pour régler la question de l'autorité parentale. Enfin, le paragraphe III concerne deux coordinations qui avaient été omises.

a été largement amputée au Sénat par un usage excessif de l'article 45 de la Constitution. En effet, des amendements relatifs à la représentation politique des Français établis hors de France

de conséquence, en commission mixte paritaire. Le bon fonctionnement du bicamérisme devrait permettre à nos deux assemblées de pouvoir débattre de l'ensemble des sujets dans des conditions similaires.

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le président de la délégation aux collectivités territoriales, en ce jeudi 12 décembre, il est minuit vingt dans la belle et paisible commune de Saint-Briac, en Ille-et-Vilaine. Vincent Denby Wilkes, son maire, rentre chez lui à pied lorsque, soudain, il se retrouve coincé par une voiture qui est montée sur le trottoir. Le conducteur en jaillit, l'insulte et le frappe violemment à trois reprises. Il réussit à s'échapper pour se réfugier dans la mairie, où il s'enferme, lumières éteintes. Son agresseur est connu en raison d'un long contentieux avec la mairie pour occupation illégale d'un terrain. Il ne sera convoqué au tribunal qu'en mai 2020. C'est à Vincent Denby Wilkes, à tous les élus victimes d'agressions que je pense ce soir, alors que nous allons voter le projet de loi Engagement et proximité destiné, entre autres dispositions, à renforcer la sécurité et la protection des maires. Le maire incarne la République et ses valeurs. Il en est le coeur, celui dont Erik Orsenna dit qu'il « répare les vivants ». Frapper un maire, c'est toucher à la République, et c'est inacceptable ! Nous devons à ces élus agressés, à tous les élus locaux

il reprend nombre de propositions majeures du Sénat sur la place essentielle de la commune au sein du bloc local. En effet, c'est le maire qui reste, pour nos concitoyens, le responsable et le comptable des décisions. conférence obligatoire des maires, au droit à l'information de tous les conseillers municipaux sur les affaires communautaires, à l'approbation du pacte de gouvernance communautaire par les conseils municipaux, à la subdélégation de la mise en oeuvre des compétences « eau et assainissement aux communes qui le demandent. Si le Sénat a confirmé la pertinence et la simplicité d'un transfert facultatif aux intercommunalités, l'Assemblée nationale a maintenu son humeur contrariée sur cette version. la solution retenue, un peu sophistiquée, doit permettre de répondre aux irritations exprimées par de nombreux élus. L'intercommunalité est une valeur ajoutée pour beaucoup de nos territoires. C'est parce qu'ici, au Sénat, nous croyons à la pertinence d'une intercommunalité de coopération que nous avons privilégié la capacité d'initiative, le sur mesure, et donc l'agilité, si nécessaire à la diversité de nos territoires. Permettre plutôt que contraindre est la leçon que nous devrions tous tirer de la loi NOTRe, qui a corseté et voulu, en quelque sorte, mettre au pas une France des territoires si pétillante d'initiatives locales. Monsieur le ministre, nous avons, avec ce texte, emprunté la voie de la différenciation de manière peu osée et un peu timide, toutefois. Je souhaite que le futur projet de loi « 3D » reprenne des propositions allantes et novatrices du du Sénat qui n'ont pas pu trouver place dans ce texte. La liberté et le sur mesure, ce n'est pas l'anarchie ; c'est le chemin de la confiance et de la responsabilité, donc de la réussite de tous les territoires dans leur diversité. Je conclurai en regrettant en regrettant que l'introduction par le Sénat de la parité dans les exécutifs communautaires, qui sont souvent des déserts féminins, n'ait pas été retenue. je salue la sagesse de l'Assemblée nationale, qui a accepté d'engager une réflexion commune et concertée avec les associations d'élus pour améliorer la parité dans l'ensemble du bloc local. Ici, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, attendre n'est pas renoncer, mais s'engager à légiférer avec plus de pertinence. Je veux remercier M. le ministre du dialogue

corapporteur de ce texte. Je salue l'engagement intense et la qualité du travail des administrateurs du Sénat. Enfin, je salue très sincèrement l'écoute toujours constructive de Bruno Questel, rapporteur du texte à l'Assemblée Ah oui ! Mes chers collègues, l'année 2019 s'achève sur un vote qui, je n'en doute pas, honorera le Parlement. Nous avons su dépasser nos différences, sans compromission, en faveur de ceux et de celles qui, jour après jour, avec générosité et modestie, servent la République. La parole est à M.

Première évolution : le texte va permettre de redonner du souffle à cette France communale à laquelle nous sommes toutes et tous attachés ici, en permettant de mettre-

entravé la ou les responsabilités de celles et de ceux qui font vivre le coeur de la démocratie locale, à savoir les élus. Nous souhaitions en effet que le texte puisse remettre

d'avoir cru en ce texte, d'avoir permis qu'il puisse aboutir lors de la commission mixte paritaire. Si nous avons eu, parfois, des débats un peu vifs avec nos collègues de l'Assemblée nationale, je veux, à mon tour, rendre hommage à notre collègue Bruno Questel,

les conditions d'exercice des mandats locaux. Beaucoup d'autres mesures viendront trouver ici une concrétisation pour le bien commun, pour le bien de nos communes et de celles et de ceux qui font vivre la démocratie. Merci à chacune et à chacun d'entre vous

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la délégation aux collectivités territoriales- cher Jean-Marie Bockel -, mesdames, messieurs les sénateurs,

et, d'autre part, monsieur le président de la commission des lois, nous avons eu un bicamérisme très performant, avec une qualité de travail assez remarquable entre les deux chambres. Je crois pouvoir le dire au nom du Gouvernement. Sachez

cette concurrence saine et très républicaine entre les valeurs de liberté et d'égalité a largement guidé nos débats, faisant parfois exploser toute forme de clivage au sein des groupes politiques. Même moi, d'ailleurs, j'ai pu être amené

Je le dis très clairement et très calmement, sur les indemnités, sujet délicat et complexe soumis à toutes les démagogies de celles et ceux qui veulent remettre en cause notre modèle démocratique, notamment la démocratie représentative,

opérationnelles, concrètes à nos collègues élus locaux pour mieux les protéger, mieux les défendre sur le terrain. Cela n'élude pas la nécessaire application des règles pénales et des poursuites judiciaires en la matière, mais, au moins, sur le terrain de la protection et de la prévention, nous avons avancé.

donner des moyens à celles et ceux qui veulent s'engager pour leurs concitoyens à quelques semaines des élections municipales. Un an après la crise dite des « gilets jaunes », voir réhabilité l'élu municipal dans son engagement, de la Ville de Paris jusqu'à la plus petite des communes de France, est quelque chose qui va dans le bon sens. C'est ça, faire Nation ! C'est ça, célébrer notre République ! La parole

ainsi que mon collègue Jérôme Durain l'avait indiqué lors de son explication de vote en première lecture, nous pouvons reconnaître au projet de loi Engagement et proximité quelques vertus.

En effet, l'un des sujets centraux devait être celui de la démocratisation des fonctions électives. Le « statut digne de ce nom », annoncé par le Président de la République, restera en deçà, malgré quelques mesures incrémentales qui

De ce volet « proximité », les sénatrices et sénateurs socialistes retirent néanmoins des points de satisfaction. Comme l'a dit le président Gérard Larcher, nous pouvons tous être des militants de l'intercommunalité, mais

En matière de participation citoyenne, l'Assemblée nationale a rétabli les conseils de développement, ce qui est une bonne chose. Je tiens par ailleurs à remercier M. le ministre d'avoir honoré son engagement quant à la possibilité de faire porter par le conseil de développement du PETR

Sur le plan des compétences, notre groupe se félicite de la généralisation de la tarification sociale de l'eau. Malheureusement, elle ne sera pas financée par l'État, contrairement aux engagements du Premier ministre aux Assises de l'eau et aux conclusions de ces mêmes assises. Si un compromis a pu être trouvé en matière d'eau et d'assainissement, il est regrettable que la compétence « tourisme » ait été remise en cause. Cela risque de compromettre des travaux d'harmonisation, notamment en termes financiers et humains, qui ont eu lieu localement dans de nombreux territoires. En matière de pouvoir de police, les nouvelles responsabilités données aux maires étaient nécessaires.

mais elles ne répondent que partiellement à la crise des vocations et, plus globalement, au manque de démocratisation du mandat local. On le sait depuis longtemps, la propension à s'engager dans la vie politique varie en fonction des caractéristiques sociales des individus. En outre, on observe une tendance à l'auto-reproduction des élus et à la perpétuation de certains d'entre eux dans le temps. Si l'on conjugue tous ces aspects sociaux avec l'incomplétude actuelle de la

Je tiens à saluer certaines avancées, notamment la revalorisation partielle du régime indemnitaire, même si les villes moyennes ne sont toujours pas concernées, le maintien des indemnités de fonction des exécutifs des syndicats, mesure que nous avions défendue, le droit à suspension du contrat de travail et à réintégration, les mesures d'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie démocratique locale, la protection fonctionnelle des maires et adjoints. ces avancées ne vont pas sans regret. Je pense à la suppression du statut de salarié protégé ou encore au financement de la revalorisation de la dotation particulière élu local, par la ponction de deux dotations perçues par les régions et les départements. en matière de formation, nous serons attentifs à l'ordonnance à venir et lirons le rapport de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection

On soulignera néanmoins que le remplacement d'un adjoint démissionnaire par un adjoint de même sexe a tout de même été instauré. C'est heureux ! Nous avions d'ailleurs soulevé cette problématique, et je tiens, monsieur le ministre, à

Le mandat de nos 600 000 élus municipaux prendra bientôt fin. Pour la moitié de nos maires actuels, ce mandat sera leur dernier. Plus de 50 % d'entre eux ne souhaitent pas se représenter en mars 2020, chiffre symbolique qui montre l'ampleur de la crise démocratique qui fait rage au coeur de nos villes et de nos villages. Ici, au Sénat, chambre des collectivités territoriales, ce chiffre nous inquiète, mais ne nous étonne guère. Au fil de nos déplacements et de nos rencontres avec des édiles en leur mairie, nous sommes témoins jour après jour de leur difficulté à poursuivre leur engagement local au service de leurs administrés. Si l'écharpe tricolore de l'élu préféré des Français est de plus en plus lourde à porter, c'est aussi notre modèle communal et notre démocratie locale qui sont en difficulté. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation des plus paradoxales : les maires sont, aux yeux de leurs administrés, responsables de tous les maux de leur cité. Or, le plus souvent, ils ne sont même plus compétents pour les soulager. ces élus du quotidien et de la proximité se sont retrouvés noyés au sein de grands ensembles, freinés par des procédures administratives de plus en plus complexes, dans un cadre financier chaque année plus contraint. Aussi, monsieur le ministre, l'annonce de votre projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a-t-il suscité beaucoup d'espoirs. Les objectifs affichés par le Gouvernement étaient ambitieux redonner des libertés locales à nos élus, lever les freins à l'engagement municipal, renforcer la cohésion de nos territoires et préserver une dynamique démocratique au coeur de nos villages. Or la montagne a accouché d'une souris, si j'ose dire. Le travail du Sénat a été à la hauteur de ces enjeux, comme l'ont notamment montré les 1 000 amendements déposés sur ce texte lors de son examen par la chambre haute. Les nombreuses heures de débats sur le couple commune-intercommunalité, sur la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales, sur le statut de l'élu local, sur la parité, sur la formation des élus, sur leur indemnisation et sur leur sécurité ont démontré les priorités incontournables que devait exprimer ce texte. C'est pourquoi nous regrettons que, malgré les frustrations générées par la loi NOTRe au sein de nos mairies, malgré cet objectif commun de « conforter chaque maire dans son intercommunalité », seules des possibilités d'adaptations ou d'assouplissements, sous contrôle de l'EPCI, aient été finalement retenues. C'est l'occasion de saluer l'excellent travail de nos rapporteurs de la commission des lois, qui s'étaient notamment attaqués au coeur du problème en proposant un transfert de compétences « à la carte Le texte du Sénat supprimait également le transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » dans les communautés de communes et les agglomérations, ce que prônait le RDSE. Nous regrettons donc que ces modifications n'aient pas été retenues par l'Assemblée nationale, puis par la commission mixte paritaire. Si ce texte peut répondre à certaines situations de blocage, concrètes, par un peu de souplesse, il ne peut prétendre à lui seul revaloriser la fonction de maire, faciliter l'exercice de son mandat et susciter de nouvelles vocations pour un engagement local. Le groupe du RDSE a joué le jeu du pragmatisme en formulant différentes propositions sur ce texte, directement issues de remontées de terrain, sans pour autant attendre la présentation du projet loi dit « 3D »- décentralisation, différenciation et déconcentration -et du projet de loi sur la sécurité locale. C'est par exemple une situation rencontrée par le maire de Salles, en Gironde, qui a motivé la création d'un droit d'information pour les maires lorsqu'une demande d'autorisation de défrichement est déposée auprès de l'autorité compétente de l'État par un des administrés de sa commune. Nous nous réjouissons que cette proposition du RDSE ait été adoptée dans la version du texte issue de la commission mixte paritaire. C'est aussi l'exemple du médiateur territorial de la ville de Bordeaux qui a inspiré la proposition de loi de Nathalie Delattre, permettant de faire prospérer un mode de règlement de conflit à l'amiable. La médiation territoriale permettra, nous en sommes convaincus, de faciliter ou de réinstaurer le dialogue entre les collectivités et leurs habitants. C'est un outil de proximité, innovant, à l'image des élus locaux et au service du bien vivre ensemble. Au nom de ma collègue et de mon groupe, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir encouragé cette proposition de loi. C'est encore par ses contacts permanents avec les élus locaux qu'Éric Gold a proposé et fait adopter l'ouverture du système d'équivalence universitaire à la valorisation de l'expérience acquise au cours des mandats, pour faciliter la reconversion des élus locaux. Nous déplorons néanmoins que certaines propositions n'aient pas reçu l'aval du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, par exemple la création d'un droit de timbre en matière d'autorisation et de déclaration d'urbanisme. Je suis d'accord ! Moi aussi et M. le président de la commission des lois, cette mesure n'a rien d'un nouvel impôt : elle constitue une simple compensation financière pour nos municipalités. compte tenu du contexte- politiques de décentralisation, encadrement de la commande publique, développement de politiques d'achat -, nous avions proposé de prévoir une indemnité spécifique pour les membres siégeant aux séances de commission d'appel d'offres et de commission de délégation de service public. Adoptée au Sénat, cette mesure a malheureusement été supprimée au cours de la navette parlementaire. Malgré des déceptions et des frustrations, notre groupe votera en faveur de ce projet de loi, dotant les maires d'une boîte à outils de secours dans l'attente d'une véritable refondation de l'édifice. La parole

monsieur le ministre, mes chers collègues, en première lecture, les apports du Sénat ont permis une amélioration du texte initial par l'intelligibilité que les sénateurs peuvent avoir des besoins des élus locaux. Je tiens ici à saluer le travail de la commission des lois, de son président et des deux rapporteurs, qui a permis de prendre en compte un certain nombre de réalités vécues et d'apporter des réponses et des solutions. Cependant, nous regrettons que les députés LREM aient détricoté dans un premier temps le texte, montrant à cette occasion leur manque de compréhension du terrain local et des enjeux du quotidien des maires.

Des avancées permettront de faire respirer les communes et leurs élus, dans leurs relations avec les EPCI comme dans leur travail au quotidien : suppression de la catégorie des compétences optionnelles, la facilitation de la répartition des compétences, l'augmentation automatique des indemnités, l'incitation à la tarification sociale de l'eau, etc.

Finalement, au lieu d'aller vers la simplicité, si chère à certains, le texte propose une redélégation afin d'en affirmer le caractère intercommunal. Il faudra suivre à terme les incidences de cette décision dans le rapport des communes au sein même de leur intercommunalité.

des nouveaux pouvoirs de police des maires et des forces de police municipale. Il ne faudrait pas donner le sentiment que les maires seraient les seuls responsables de la sécurité ou de la tranquillité publique- chacun utilisera l'expression qui lui agrée. effet aujourd'hui la préoccupation première des habitants pour les prochaines élections municipales. Rappelons que la question de la sécurité est et doit rester une compétence régalienne. Or, au vu du déploiement- du non-déploiement, devrais-je dire -de la gendarmerie comme de la police, de la difficulté à satisfaire tous les postes, des fermetures et restructurations subies depuis de nombreuses années, les maires se retrouvent souvent seuls à répondre à ce besoin de sécurité exigé par nos concitoyens. des conditions de travail et du quotidien des élus locaux. Nous sommes pour les mesures prévues, telles qu'elles sont inscrites à l'issue de la commission mixte paritaire. nous ne pouvons qu'être inquiets, puisque la pression financière exercée aujourd'hui sur les collectivités peut en limiter l'effectivité. Enfin, la Enfin, la démocratie locale doit être développée par de nouveaux outils et les services publics qui font le lien entre les citoyens et le politique. Or la liste de ceux qui disparaissent est nombreuse : finances publiques, trains, hôpitaux, plus largement la présence territoriale de l'État dans nos départements. À ce rythme-là, dans quelques mois, il sera plus rapide de citer les seuls services publics restant dans nos territoires. Monsieur le ministre, au quotidien, c'est à tout cela

être élu, oui, mais pour quoi faire demain ? Quels moyens pour répondre aux besoins des populations ? Certes, ce texte marque un coup d'arrêt à la mécanique décriée lancée par la loi NOTRe. Il signifie que la mobilisation et les craintes des élus commencent enfin à être entendues, bien que l'examen du texte par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale laisse planer le doute quant à cette finalité. La crise de l'engagement a besoin d'une véritable réponse et les collectivités territoriales doivent être revitalisées, en termes de services publics, en termes humains, en termes de démocratie locale et plurielle. Nous nous abstiendrons sur ce texte.

retenue. Elle consiste à relever de manière raisonnable le montant maximal des indemnités des élus des communes de moins de 3 500 habitants, tout en permettant au maire de solliciter une réduction de son indemnité, s'il le désire. Les maires et élus de ces communes seront augmentés automatiquement, selon trois tranches, ce qui évite de solliciter l'augmentation au conseil municipal comme le prévoyait la version de l'Assemblée nationale 50 % de plus pour les élus des communes de moins de 500 habitants, 30 % de plus pour les communes de 500 à 999 habitants et 20 % de plus pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants. Je suis heureux que ce texte valorise ainsi le rôle des élus locaux dans notre démocratie. En effet, chez les élus, un sentiment latent de dépossession s'est installé. Successivement, ils ont dû affronter les baisses de dotations de l'État, qui ont affecté toutes les collectivités de manière indistincte et non concertée, concertée, puis la marche forcée vers les grandes intercommunalités et les grandes régions. Je me réjouis donc tout particulièrement que ce projet de loi entende accompagner ceux qui s'engagent pour la collectivité, en améliorant les conditions d'exercice des mandats locaux. Je me félicite également que ce texte étende les libertés locales, conforte le rôle du maire pour trouver un meilleur équilibre avec son intercommunalité, simplifie le quotidien des élus locaux et adapte mieux certaines règles ou seuils aux réalités territoriales. l'ensemble des dispositions de ce texte constituent un progrès pour que les communes et communautés de communes jouent à nouveau un rôle essentiel dans l'histoire de notre démocratie, mais nous espérons que le projet de loi Engagement et proximité sera utilement

Françoise Gatel et Mathieu Darnaud. Je salue également l'immense travail accompli par les élus locaux, au premier rang desquels les maires, qui sont au plus près des citoyens, de leurs demandes, de leurs encouragements ou de leurs récriminations. Je pense aussi aux maires des petites communes rurales, qui ne comptent pas leur temps et sacrifient bien souvent une partie de leur vie professionnelle et familiale à leur mandat. Je suis aussi élu local, je me sens proche de leurs inquiétudes et de leurs interrogations. Monsieur le ministre, mes chers collègues, particulièrement attentif aux préoccupations exprimées par les collectivités territoriales,

soit sur le point d'être définitivement adopté, puisqu'il contient de nombreuses mesures attendues par les élus, je pense que la procédure accélérée aurait pu être écartée

pour les collectivités territoriales et au vu des nombreuses dispositions additionnelles adoptées sans étude d'impact approfondie, je trouve que notre travail de législateur s'est fait avec une grande qualité, mais à marche forcée. Espérons que nous ne regretterons pas dans quelques mois de ne pas avoir donné un peu plus de temps au Parlement pour nous assurer de la justesse et de l'opportunité de toutes les dispositions que nous nous apprêtons à adopter. Sur le fond, je tiens à rappeler que, dans la préparation de ce texte, le Gouvernement s'est largement inspiré de nombreux travaux du Sénat, notamment ceux de

commission mixte paritaire préserve de nombreux apports du Sénat. Ainsi, dans le cadre de l'élaboration du pacte de gouvernance, le Sénat a tenu à ce qu'il ne puisse être adopté qu'après avis des conseils municipaux des communes membres. Par ailleurs, un amendement du groupe Union Centriste a rendu obligatoire la création d'une conférence des maires au sein de l'ensemble des EPCI. C'était d'ailleurs une demande assez large. Le Sénat a également souhaité que ce texte de simplification soit l'occasion de supprimer la catégorie des compétences optionnelles des intercommunalités. Demain, les intercommunalités conserveront les compétences obligatoires aujourd'hui définies par la loi, auxquelles pourront s'ajouter des compétences facultatives. Cette mesure de clarification a été efficacement défendue par les représentants de la commission des lois en commission mixte

aux communes et aux syndicats. Le Sénat a également introduit une disposition prévoyant que la caducité des plans d'occupation des sols, prévue au 31 décembre 2019, soit repoussée d'un an

pour faire respecter leurs arrêtés de police et pour garantir leur protection contre les violences ou les incivilités. Sans doute faudra-t-il en évaluer l'efficacité après quelques années de mise en oeuvre, soit pour les simplifier, soit pour les renforcer. Le retour d'expérience est nécessaire. Sur les dispositions relatives aux indemnités des élus des communes de moins de 3 500 habitants, la commission mixte paritaire a retenu la proposition adoptée par le Sénat en première lecture, qui est un système plus simple et plus lisible que le dispositif baroque adopté par nos collègues députés. Sur le régime indemnitaire des présidents et des vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes, le Sénat a supprimé une disposition inopportune de la loi NOTRe et ainsi maintenu leurs indemnités de fonction. En confirmant cette disposition, la commission mixte paritaire

des évolutions inéluctables et positives. Je tiens une fois encore à saluer l'excellence du travail de nos rapporteurs, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel,

Ils peuvent être fiers du travail accompli et du texte qu'ils soumettent au Sénat aujourd'hui. C'est une étape utile pour la simplification du travail des élus, un signal politique de considération en direction des élus locaux, qui forment le tissu civique de notre pays, et une amélioration concrète de leurs conditions d'action. C'est aussi une réponse à la crise des vocations, qui est devenue

En effet, la situation laissée par la loi NOTRe sur le terrain s'est révélée pour le moins inadaptée, face à l'exercice quotidien du mandat des élus, toujours plus complexe et difficile. C'est la raison pour laquelle le Sénat a rapidement pris l'initiative : il a présenté des propositions de loi, des rapports d'information et a interpellé le Gouvernement. Le travail réalisé au Sénat a porté ses fruits. Dès la version initiale du projet de loi Engagement et proximité, la marque de notre assemblée était visible dans un certain nombre de ses propositions, révélant l'intérêt que leur portait le Gouvernement. Certains volets du projet d'origine

Aujourd'hui, l'examen de ce projet de loi arrive à son terme. La commission mixte paritaire du 11 décembre dernier a abouti à un texte de compromis reprenant nombre des avancées sénatoriales. Je tiens à cette occasion à saluer les rapporteurs Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, qui ont accompli un travail remarquable en commission, dans notre hémicycle ainsi que dans le cadre de la négociation avec les députés, négociation ardue, mais réussie. Venons-en au texte lui-même. On y devine désormais encore plus aisément la marque de l'expertise sénatoriale. En particulier, le Sénat a porté une vision renouvelée de l'intercommunalité. Il a réaffirmé la place centrale de la commune et des élus communaux, en systématisant les conférences des maires ou encore en renforçant le poids des communes dans les CDCI. Il a réintroduit une dose de simplicité, par la suppression des compétences optionnelles. Il a amélioré l'information des élus communaux sur les affaires intercommunales. notre conviction est que la commune est la cellule de base de la République. Comme le souligne régulièrement notre président Gérard Larcher, elle est « la petite République dans la grande ». À ce titre, elle doit pouvoir avoir les moyens de de jouer ce rôle. Ces moyens impliquent aussi une consolidation des pouvoirs de police des maires et une meilleure coordination de l'action des forces de sécurité de l'État et des collectivités. C'était notre objectif au moment de la présentation du plan d'action pour une plus grande sécurité des maires, qui a contribué à irriguer les travaux du Sénat sur votre projet de loi, monsieur le ministre. Ici aussi, ce sont bien les remontées du terrain qui nous ont guidés. Les maires nous ont fait part de leur lassitude face à une certaine impuissance, par exemple lorsqu'ils ne sont pas informés de l'aboutissement des procédures qu'ils lancent. Ils ont aussi partagé avec nous leur inquiétude face aux risques juridiques pesant sur eux. C'est vrai ! Nous avons choisi d'offrir des solutions : une meilleure information des maires par le procureur, des pouvoirs de police plus étendus pour les maires, policiers municipaux et gardes champêtres, une consolidation du cadre des conventions de coordination entre police municipale et forces de sécurité de l'État, une assurance juridique renforcée. Enfin, pour lutter contre le mal-être des élus, le projet de loi vise à la fois à simplifier leur quotidien et à mieux reconnaître leurs droits. L'ambition est de taille. Sans prétendre révolutionner la vie des collectivités, le texte final constitue,

pourront tout particulièrement bénéficier de ces hausses d'indemnités. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, les maires pourront toujours demander d'obtenir un montant d'indemnités inférieur s'ils le jugent préférable. Au-delà de cette mesure particulière, défendue par notre rapporteur Mathieu Darnaud, le texte comprend d'autres avancées proposées par le Sénat, comme des dispositions destinées à favoriser l'accès aux mandats électifs des personnes souffrant d'un handicap, à assurer une meilleure formation des élus ou encore à préserver les indemnités des présidents et des vice-présidents de certains syndicats, lesquelles auraient été supprimées par la loi actuelle. Après la transmission du texte ainsi enrichi à l'Assemblée nationale, une trentaine d'articles ont été adoptés sans modifications par les députés. Nous saluons leur réceptivité aux idées du Sénat. Nous avions cependant aussi observé avec une certaine inquiétude la suppression, dès l'examen du texte en commission, d'un grand nombre des apports les plus importants de notre assemblée. Certains ont fini par par être curieusement restaurés en séance publique, parfois même sur l'initiative du Gouvernement. Je m'arrêterai quelques instants sur l'un des apports de l'Assemblée nationale : l'article portant sur l'application de la parité dans les petites communes. Permettez-moi d'abord de rappeler que la question de la parité n'avait pas été négligée par le Sénat. Nos rapporteurs avaient proposé un dispositif destiné à garantir une plus grande représentation des femmes dans les organes délibérants des EPCI. Les députés l'ont supprimé, préférant instaurer un scrutin de liste paritaire dans les communes de plus de 500 habitants, contre 1 000 aujourd'hui. Cette mesure, qui part d'une intention louable -renforcer la place des femmes parmi les élus

Je salue donc le choix qui a été fait en commission mixte paritaire de ne pas inclure cette disposition dans le texte final, afin de prendre le temps de trouver d'autres solutions, moins dommageables pour la vie démocratique de nos communes. La question de la représentation des femmes au sein des instances décisionnelles locales est trop importante pour que nous puissions nous permettre d'en passer par des dispositifs aux effets aussi ambigus. Certes, toutes nos positions n'ont pas été reprises. En dépit de certains progrès, nous n'avons réussi à obtenir ni la fin du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement », ni la possibilité de transférer des compétences « à la carte ». La question des accords locaux de répartition des sièges demeure ouverte et devra tôt ou tard être traitée. Des mesures aux effets limités, comme la célébration des mariages hors de la mairie, ont également disparu de la version finale du texte. Enfin, le Gouvernement et les députés ont souhaité écarter un certain nombre de points, en particulier ceux relevant de près ou de loin de la différenciation. Ils ont justifié leur décision par l'arrivée prochaine du projet de loi « 3D ». Nous en prenons bonne note, monsieur le ministre, mais on nous dit que ce

ainsi que d'autres, car personne ici n'imagine que le présent projet de loi a permis de faire le tour des problématiques territoriales. Apporter des correctifs aux irritants de la loi NOTRe est louable, mais apporter des solutions durables et structurantes est préférable

la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale,